Monsieur le ministre, mes chers collègues, cher Jean-Claude Guibal, chères Géraldine et Céline, c'est avec une profonde tristesse que nous avons appris, le 24 septembre dernier, la disparition de notre collègue Colette Giudicelli, sénateur des Alpes-Maritimes depuis 2008. Mme Dominique Estrosi Sassone, elle-même sénateur des Alpes-Maritimes, a représenté le Sénat aux obsèques, célébrées le 28 septembre en la basilique Saint-Michel-Archange de Menton, en présence du Prince souverain de Monaco, du préfet des Alpes-Maritimes et de nombreux collègues élus du département, obsèques qui ont rassemblé une foule de Mentonnais, venus témoigner de leur gratitude et de leur attachement à une femme dynamique et passionnée, qui a consacré une grande partie de sa vie à ses concitoyens et à la ville de son coeur. Première femme dans l'histoire parlementaire à être élue sénateur des Alpes-Maritimes en 2008, réélue en 2014, elle siégeait dans notre hémicycle depuis près de douze ans. Nous garderons d'elle le souvenir d'une collègue fortement impliquée dans les travaux parlementaires concernant, notamment, les questions sociales et la santé, mais aussi l'image d'une élue de terrain devenue une figure emblématique du pays mentonnais, une personnalité attachante au caractère bien trempé. Colette Giudicelli fut, dès sa jeunesse et tout au long de sa vie, une femme de convictions, fidèle à ses engagements pour défendre ses idées et ce qu'elle croyait juste. Née le 24 novembre 1943 à Alger, elle était issue d'un milieu modeste : son père était ouvrier et président de l'Association des Corses d'Alger sa mère était femme au foyer. Ses grands-parents paternels, agriculteurs originaires de Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio, étaient venus s'installer en Algérie. À Alger, Colette Giudicelli résidait dans le quartier de Belcourt, où toutes les communautés se mélangeaient, chrétiens, musulmans et juifs vivant alors dans une réelle harmonie. Elle garda toujours un merveilleux souvenir de cette convivialité. À l'issue de ses études secondaires au lycée Delacroix, elle poursuivit des études de philosophie et de pharmacie. Amoureuse de la langue russe, elle apprit à la parler. Après l'indépendance de l'Algérie, sa famille vint s'établir à Lyon, puis Colette Giudicelli finit par trouver à Menton un peu de l'atmosphère méditerranéenne qui lui manquait tant. Animée par l'envie de se mettre au service des autres, elle s'engagea très tôt au sein du secteur associatif, tant éducatif que social. Ainsi, elle devint représentante des parents d'élèves de l'institution Saint-Joseph, établissement d'enseignement accueillant les enfants de la maternelle à la terminale, puis, pendant de nombreuses années, cette femme de coeur assura avec une attention sans faille sa fonction de présidente du conseil d'administration de l'institut médico-éducatif Bariquand-Alphand, qui accueille des enfants souffrant de handicaps mentaux. Elle s'est également beaucoup impliquée dans l'association caritative mentonnaise Les Coeurs de Campanin, qui fournit une aide alimentaire aux personnes en difficulté. C'est en suivant Jean-Claude Guibal, qui allait devenir son époux et dont elle a été la première adjointe à la mairie de Menton pendant vingt ans, que Colette s'était engagée en politique, alors que rien, dans ses goûts et ses affinités, ne la prédestinait à cet engagement. Elle accéda ainsi pour la première fois à des fonctions politiques en étant élue conseillère municipale de Menton en 1989, auprès de celui qui est resté à ses côtés jusque dans les dernières épreuves. Ils formèrent ensuite, pendant des années, un « couple » de parlementaires, elle comme sénateur et lui comme député. Quelques mois seulement après son élection au conseil municipal de Menton, Colette Giudicelli devint première adjointe au maire, chargée de l'administration générale, des finances et du personnel, fonction qu'elle exerça avec ténacité et dévouement durant deux décennies. Après avoir siégé au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur de 1998 à 2001, elle fut élue conseillère générale du canton de Menton-Est à partir de 2001, puis élue départementale du canton de Menton tout entier après 2015. Là encore, elle exerça des responsabilités exécutives : comme vice-présidente du conseil général, puis du conseil départemental, et ce de 2001 à 2017, elle défendit avec compétence et pugnacité les dossiers concernant les finances, l'administration générale et le personnel. Depuis 2002, elle était également devenue vice-présidente de la communauté d'agglomération de la Riviera française. Lorsqu'elle fit son entrée au Sénat en 2008, Colette Giudicelli, fidèle à l'engagement social qui avait toujours été le sien, souhaita tout naturellement rejoindre la commission des affaires sociales. Aspirant à contribuer à ce « que à ce « que la législation améliore le sort des plus démunis », elle consacra son ardeur au travail et sa force de caractère aux travaux parlementaires dans les secteurs de la santé, du handicap et du logement. Dès 2010, elle s'investit tout particulièrement dans une mission de contrôle budgétaire sur la mise en place du revenu de solidarité active. Animée par le souci de favoriser plus de justice et d'équité, elle prit l'initiative de déposer, en 2014, une proposition de loi visant à modifier les conditions d'attribution des logements sociaux, afin de promouvoir la mobilité au sein du parc locatif social. Son souhait de libérer la parole des médecins pour faciliter le secours aux enfants maltraités fut à l'origine de l'adoption de la loi du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé. La proposition de loi qu'elle avait déposée pour protéger l'ensemble des médecins des poursuites qui pourraient leur être intentées en cas de signalement et, partant, renforcer et encourager leur mission de protection des mineurs fut en effet adoptée à l'unanimité de tous les groupes, au Sénat puis à l'Assemblée nationale. Colette Giudicelli apporta également une contribution aux travaux législatifs de la commission des affaires sociales, comme rapporteur d'un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, notamment en matière de santé, santé, en 2011, puis du projet de loi de financement de la sécurité sociale, pour le secteur médico-social, en 2015. Toujours dans le domaine de la santé, elle fut en outre l'auteur d'un rapport d'information sur la prévention du suicide. Son engagement en faveur des handicapés fut consacré par sa nomination, en 2014, comme membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Sa curiosité d'esprit Sa curiosité d'esprit la conduisit par ailleurs à participer à de très nombreuses structures sénatoriales temporaires, essentiellement dans le domaine social. Comme présidente du groupe interparlementaire d'amitié France-Monaco, Colette Giudicelli s'est attachée à développer les relations avec la Principauté monégasque, si proche et si chère à son J'ai le souvenir de ma visite officielle, les 15 et 16 mars 2019, à la Principauté de Monaco, en présence du Prince souverain Albert II. Colette était là, bien que souffrante, lorsque j'ai les insignes de chevalier de la Légion d'honneur au président du Conseil national monégasque, et j'étais heureux de cette rencontre entre les deux chambres

Je célébrais alors la communauté de destin unissant nos deux pays, reposant sur une coopération étroite dans les domaines économique, fiscal, scientifique et culturel. Colette y est restée fidèle tout au long de son engagement. Sa dernière intervention en séance publique, avant que l'évolution de son état de santé la contraigne malheureusement à devoir renoncer à se rendre au Sénat, fut une ultime démonstration de son attention permanente aux questions de santé elle tenait ce jour-là, monsieur le ministre, à alerter le Gouvernement au sujet des émanations dangereuses provenant d'huiles de moteur qui peuvent contaminer le système d'alimentation en air des avions, au risque de provoquer de graves perturbations neurologiques. Je me souviens aussi d'avoir accueilli Colette Giudicelli, dans les salons de la présidence du Sénat, lors de la cérémonie au cours de laquelle Christian Estrosi, alors ministre de l'industrie et maire de Nice, lui avait remis les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Il avait à cette occasion salué une femme pour qui « le sens du devoir [était] toujours passé avant le goût des honneurs ». En réponse, elle s'était alors dite « fière de pouvoir affirmer avoir toujours eu pour seul objectif le bien public et la volonté d'être au service de ses concitoyens Elle maîtrisait ses dossiers et avait à coeur de poursuivre ses engagements. Reconnue pour son dévouement, notamment auprès des personnes en difficulté sociale, c'était cette élue de terrain que j'ai décrite. Elle avait aussi réussi à conjuguer son action au service du bien commun avec une attention particulière à l'égard de ses enfants et de ses petits-enfants. Je tiens à rendre hommage à ses qualités humaines : courage force de caractère, alliés à la bienveillance, la générosité et la gentillesse. À ses anciens collègues de la commission des affaires sociales

j'exprime ma sympathie, comme je le fais à l'égard de ses amis du groupe Les Républicains, qui l'ont vue partir quelques jours avant le renouvellement sénatorial. À Jean-Claude Guibal, maire de Menton, que je salue tout particulièrement, à ses filles Céline et Géraldine, ici présentes, à l'ensemble de sa famille et de ses proches, à tous ceux qui ont partagé ses engagements, à Menton, dans la vie, et ici, au Sénat, je souhaite redire la part que le Sénat prend à leur deuil.

tout aussi enracinée, libre et forte qu'ouverte sur le monde et ses horizons, Colette Giudicelli était à l'image de la ville de Menton, qu'elle aimait passionnément. Née à Alger le 24 novembre 1943, issue d'une famille aux origines modestes, elle portait en elle quelque chose des secrets de la Méditerranée. Sans doute cette façon simple et instinctive de se sentir ancrée dans une terre et de vivre une identité plurielle, chaleureuse, mais franche et directe dans son rapport à l'autre, cet autre qui nous ressemble, malgré ses différences. Cette volonté d'aller vers l'autre, encore et toujours, Colette Giudicelli savait la transmettre d'un regard, d'un sourire ou d'une poignée de main à celles et ceux qui la croisaient dans les rues de sa ville. Il s'agissait du sens même de son engagement politique, de ce qu'elle était profondément. À Menton, nombreux sont venus s'en souvenir dans le hall d'entrée de la mairie, en se recueillant sur sa photo, posée tout simplement sur une table de bois à côté d'une orchidée blanche. Ils se sont ainsi souvenus qu'en 1985 ils ont fait confiance à cette mère dévouée, qui s'était alors entièrement consacrée à l'éducation de ses enfants, et qu'ils ont aimé la voir prendre goût à l'action locale lors d'une campagne municipale menée aux côtés de Jean-Claude Guibal. Elle y insuffle toute son énergie, son enthousiasme et son sens de l'initiative, si bien que, en 1989, elle est l'artisan de la victoire de celui qu'elle prendra par la suite pour époux, la ville de Menton devenant le trait d'union de leur engagement. Conseillère municipale et très vite première adjointe, Colette Giudicelli fait immédiatement preuve d'une détermination et d'une énergie sans faille dans la conduite des dossiers qui lui sont confiés, à savoir l'administration générale, les finances et les quartiers, donnant d'emblée à voir les qualités qui allaient la définir tout au long de sa vie publique. En 1995, elle poursuit son action locale avec une délégation étendue à la sécurité et à la prévention de la délinquance. De nouveau élue en 2001, elle s'engagera sans compter, comme elle le faisait toujours, en prenant à bras-le-corps les questions relatives au sport, à la communication et à la promotion, ainsi qu'à la vie des quartiers. En 1998, cet engagement municipal va trouver son prolongement avec l'élection de Colette Giudicelli au conseil régional, mais aussi, et peut-être surtout, au conseil départemental des Alpes-Maritimes, mandat auquel elle était profondément attachée. Élue du canton de Menton-Est, elle était chargée de la politique de la ville, de la vie des quartiers et de l'insertion. Son bilan lui permettra d'obtenir de nouveau la confiance des habitantes et des habitants de son canton en 2011. Elle devient alors la première femme vice-présidente du conseil départemental et, sous son impulsion décisive, l'institution fait de la lutte contre les ségrégations urbaines et sociales l'une de ses priorités. La vie associative des quartiers, dont elle a la responsabilité, l'amène à s'engager dans de nombreux combats combats : la protection de l'enfance, l'alphabétisation et le soutien aux femmes dans le cadre des contrats de ville. Elle s'investit totalement pour mener à bien chaque dossier en mettant, comme elle le disait, « les mains dans le cambouis Son engagement politique, qu'elle vivait avec entièreté, ne la détournera pourtant jamais des activités associatives auxquelles elle prenait part depuis 1976 au sein des associations de parents d'élèves des écoles et collèges Saint-Joseph à Roquebrune-Cap-Martin et Maurois à Menton. Elle était en effet de toutes les manifestations, que ce soient les sorties pédagogiques, les classes vertes ou les kermesses scolaires. Celles et ceux qui ont eu à travailler avec elle dans le cadre de ses engagements publics locaux savent que Colette Giudicelli était viscéralement attachée à sa terre et qu'elle avait, par conséquent, aussi à coeur de défendre et promouvoir les Alpes-Maritimes au niveau national. C'est ainsi qu'en 2008 elle devint la première femme sénatrice de son département. Elle aimait profondément ce mandat pour ce qu'il est : celui du lien charnel à un territoire ; celui de l'authenticité et de la proximité ; celui de la confiance qui se gagne par ce qui est fait. Au Sénat, Colette Giudicelli s'est investie avec enthousiasme et efficacité à la commission des affaires sociales, dont elle a été vice-présidente. Active et engagée sur les sujets liés au social et au médico-social, comme vous l'avez rappelé, monsieur le président, à l'éducation, au handicap et au grand âge, elle voulait, au travers de chacune de ses interventions, prolonger et, au fond, amplifier l'action qu'elle menait alors au sein du département des Alpes-Maritimes. C'est dans cette logique qu'elle décidera de porter un combat décisif en faveur de la protection de l'enfance, en étant à l'origine de la loi du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé. Cette loi, qui permet de protéger l'ensemble des médecins des poursuites qui pourraient leur être intentées en cas de signalement des violences faites aux enfants, marque une étape importante et décisive en la matière. Battante, infatigable, elle s'est éteinte à la fin de son mandat de sénatrice en septembre dernier, comme pour nous dire que sa vie et son engagement au service de son territoire avaient toujours été intrinsèquement liés. À son époux, à ses filles, à ses proches, à ses anciennes et anciens collègues du Sénat, à ses amis et collègues du groupe Les Républicains, à celles et ceux qui ont été à ses côtés dans sa vie publique, aux habitantes et aux habitants des Alpes-Maritimes et, évidemment, de Menton, j'exprime, au nom du Gouvernement, nos condoléances les plus sincères et le témoignage de notre profonde sympathie.

La séance est reprise. Mes chers collègues, pour le respect des règles sanitaires, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans l'ensemble du palais, y compris pour les orateurs. Il vous est demandé de laisser un siège vide entre deux sièges occupés. J'invite chacune et chacun d'entre vous à veiller au respect des distances de sécurité. Je rappelle également que les sorties de la salle des séances devront exclusivement s'effectuer par les portes situées au pourtour de l'hémicycle. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission spéciale, cher Jean-François Longeot, mes chers collègues, je suis heureux de présenter aujourd'hui au vote de notre assemblée le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire qui s'est tenue au Sénat le 21 octobre dernier. nous sommes parvenus, députés et sénateurs, à nous accorder sur un texte qui apportera des avancées importantes à nos concitoyens. Pourtant, les conditions d'examen de ce texte étaient compliquées à plusieurs titres.

mais aussi des remords du Gouvernement, qui, par amendements, n'a eu de cesse d'alourdir la barque avec des dispositions importantes, qui ne sont ni validées par le Conseil d'État ni évaluées. Ce projet de loi est ainsi passé de 50 articles à plus de 160 examinés trop rapidement en procédure d'urgence. Ensuite, après la première lecture au Sénat au mois nous avons connu une interruption de plus de six mois due à la crise sanitaire, avant la reprise de la discussion par l'Assemblée nationale. Si nous avons malgré tout réussi à trouver un accord global, c'est sans doute grâce à une volonté partagée d'écoute et d'ouverture transpartisane entre les commissions spéciales de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je souhaite à cet

Guillaume Kasbarian, avec lequel j'ai eu des discussions franches et constructives. Cet accord porte la marque du Sénat, qui a fait prévaloir de nouveaux de nouveaux équilibres et de meilleures garanties juridiques. Je pense précisément à l'attention particulière portée aux collectivités locales, dont nous avons préservé et augmenté les compétences, qu'il s'agisse du renforcement de l'information des maires sur les projets d'installations éoliennes ou de la préservation du permis d'aménager et de l'obligation d'information dans l'exercice du droit d'initiative. Le Sénat y était très attaché : les élections

Le Sénat a également amélioré les dispositifs concernant la vente en ligne de produits pharmaceutiques et l'alimentation du dossier pharmaceutique. En première lecture, au Sénat, le sujet de la vente en ligne a constitué une question majeure sur laquelle un bon équilibre Nos collègues députés ne l'ont pas remis en cause. De même, je suis très satisfait que, sur la question de l'alimentation du dossier pharmaceutique par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et médico-sociaux, le Sénat ait retenu un dispositif qui bénéficiera à tous les patients.

Sur les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, au traitement des sols pollués ou encore les dispositions relatives à l'information et à la participation du public, nous sommes parvenus à un compromis assez équilibré, qui permet de préserver la portée du droit de l'environnement, tout en favorisant l'attractivité de nos territoires, donc les installations industrielles et la création d'emplois. L'équilibre n'était pas facile à trouver ; il a été trouvé. Nous avons également obtenu de bons compromis compromis : sur la suppression de la Commission scientifique nationale des collections, remplacée par des mécanismes visant à garantir un contrôle scientifique préalable à toute décision de déclassement sur la possibilité pour les personnes âgées résidant dans un établissement médico-social d'utiliser leur chèque énergie pour régler certaines dépenses ; sur la protection des consommateurs dans le cadre des transferts de réseaux de gaz ; sur l'extension au biogaz des souplesses administratives prévues pour l'électricité renouvelable ; et aussi sur la suppression des certificats médicaux pour l'exercice d'un sport par les mineurs.

ce dossier. Nous avons retenu la version adoptée par le Sénat, c'est-à-dire le renforcement du droit de résiliation annuelle, qui est la formule la plus sûre et dont les effets ont été évalués.

En second lieu, nous avons amélioré le dispositif introduit par l'Assemblée nationale et ayant pour objet de renforcer la procédure d'expulsion des squatteurs en limitant les cas dans lesquels le préfet peut refuser de mettre en demeure l'occupant des lieux. Il s'agit des cas où les conditions fixées par la loi ne sont pas respectées- demande incomplète, squat non attesté, etc. -ou lorsqu'un motif impérieux d'intérêt général est en jeu.

À ce titre, nous ne pouvons que déplorer le recours excessif aux ordonnances et le fait que des dispositions soient prises sans que le Parlement ait préalablement débattu au fond.

Or jamais un ministre n'a débattu au Parlement des objectifs du SNU, de sa mise en place, des moyens humains et budgétaires à mettre en oeuvre, de son calendrier. Pour ma part, la concession la plus difficile à accepter a été de retenir la rédaction de l'article 33 proposée par l'Assemblée nationale concernant les agents de droit privé de l'Office national des forêts (ONF). Ces agents nouvellement recrutés pourront ainsi verbaliser les infractions au-delà des seules infractions forestières. Je le regrette, car nous devrions tout au contraire recentrer l'action des agents sur l'entretien et la gestion de nos forêts dont nous connaissons l'état dramatique.

S'agissant de l'article 33, je me félicite en revanche de ce que l'habilitation à légiférer par ordonnance sur le conseil d'administration de l'ONF ne figure plus dans le texte final. Par ailleurs,

que je vous invite à voter le texte du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), qui résulte des travaux de la commission mixte paritaire. À ce stade, je remercie le président de la commission spéciale, Jean-François Longeot,

les arbitrages que nous avons rendus avec l'Assemblée nationale. La parole

Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs,

Sur la simplification du quotidien des Français, ce texte vise à répondre aux préoccupations des Français, qui se sont notamment exprimées pendant le grand débat national. Sur la simplification des entreprises, ce texte rassemble les propositions de la mission Kasbarian réalisée pour le groupe de travail Industrie dans le cadre de la préparation du Pacte productif. Ce texte a été conçu avant le covid et voté au début du mois de mars dernier au Sénat. La crise que nous traversons nous a montré que nous pouvions aller plus loin et nous engager plus avant dans cette simplification. Le texte a ainsi été enrichi par un travail interministériel conduisant à identifier deux types de simplifications additionnelles

Les deux premiers titres de ce projet de loi traduisent les engagements pris par le Gouvernement en matière d'organisation administrative. Le premier de ces engagements, c'est celui d'une organisation administrative plus simple et plus réactive. Vous le savez, le comité interministériel de la transformation publique prévoyait de supprimer 86 commissions consultatives sur les 394 existantes. Certaines ont une accroche législative et seront supprimées par cette loi. Cette simplification vise à fluidifier de manière significative le processus de la décision publique, bien souvent perçu comme trop lent et complexe par nos concitoyens, nos élus locaux et nos entreprises. En même temps, nous avons écouté les considérations des parlementaires et maintenu les commissions qui paraissaient essentielles. Ainsi, à la demande du Sénat, la commission mixte paritaire a maintenu la Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs Le second engagement du Gouvernement consiste à rendre les administrations plus proches et plus accessibles. Notre objectif consiste à approcher un taux de 99 % de décisions individuelles prises à l'échelon local. Une administration plus proche et plus à l'écoute de nos concitoyens, ce n'est pas qu'un impératif d'efficacité, c'est également un impératif démocratique. Les deux chambres se sont retrouvées sur ce sujet, qui a été adopté de manière consensuelle en commission mixte paritaire. Les titres III à V du projet de loi visent des simplifications pour le quotidien des Français et des entreprises. Leur objectif est de faire gagner du temps à nos concitoyens et à nos administrations, pour que ces dernières se concentrent sur les sujets ayant la plus grande importance pour les Français. Ce texte permet de simplifier les démarches administratives : faciliter la délivrance de différents documents comme les papiers d'identité ou le permis de conduire ; simplifier des démarches qui concernent nos jeunes concitoyens, que ce soit pour passer le permis de conduire ou la pratique du sport simplifier les ouvertures de livret d'épargne populaire pour nos concitoyens aux revenus les plus modestes. Nous assumons cette diversité de mesures, car ce sont précisément celles qu'attendent nos concitoyens. Cela ne fait peut-être pas la une des journaux, mais, en tout état de cause, cela facilitera leur quotidien. Par ailleurs, les travaux des deux chambres ont permis d'enrichir le texte de nouveaux axes de simplification pour protéger les Français : simplification et accélération de la procédure administrative d'expulsion en cas d'occupation illicite du domicile et renforcement des sanctions pénales anti-squat pénales anti-squat ; extension de l'utilisation des chèques énergie aux hébergements pour personnes âgées. Le projet de loi vise également à simplifier la vie de toutes les entreprises. Le premier axe concerne les procédures des implantations et extensions industrielles que le Gouvernement souhaite accélérer sans modifier de normes d'urbanisme, d'archéologie ou d'environnement. Les délais pour une décision d'autorisation sont deux fois plus longs en France qu'en Suède. Pourtant, le droit suédois est au moins aussi exigeant que le nôtre en matière d'environnement.

Pour raccourcir les délais tout en maintenant nos exigences en matière environnementale, culturelle et de droit de l'urbanisme, des « sites clés en main » ont été identifiés, pour lesquels toutes ces procédures administratives ont été menées en amont. Un projet industriel pourra ainsi démarrer sa production en quelques mois seulement. Il s'agit de créer de l'emploi sur notre territoire national. Le deuxième axe consiste à anticiper et faciliter les procédures pour accélérer le déploiement de la relance. C'est un point qui est cher au ministère de l'économie, des finances et de la relance, en particulier à Bruno Le Maire et à moi-même. Le projet de loi ASAP permet d'aller plus loin dans le partage de la valeur. Des dispositions sont prévues pour faciliter les négociations en matière d'épargne salariale et d'accord d'intéressement. Nous tirons là les enseignements de la mise en oeuvre de la loi Pacte. Le projet de loi ASAP permet également d'aller plus loin pour faciliter la commande publique, en pérennisant certains dispositifs pris pendant l'état d'urgence sanitaire et en augmentant le seuil de la commande publique sans formalité pour les travaux à 100 000 euros pendant les deux ans de la relance. Ce faisant, nous nous rapprochons de la moyenne européenne.

vous pouvez le constater : ce texte est utile et concret. Je veux ici saluer le travail de concertation et de coconstruction qui a rendu possible son adoption rapide. ce projet de loi a été peu à peu enrichi par vos apports et le débat parlementaire. Je tiens à cet égard à souligner le travail accompli par les deux chambres, plus particulièrement en ce jour par le Sénat. Votre esprit d'exigence et de dialogue a permis de faire avancer ce texte, afin qu'il réponde aux attentes formulées par nos concitoyens.

Même si les rédactions ont pu évoluer, les simplifications de l'administration et celles pour les implantations industrielles se sont révélées consensuelles. C'est la preuve que ces mesures ont du sens pour nous tous, pour favoriser la localisation d'activités et d'emplois dans nos territoires sans en rabattre sur nos standards environnementaux. maintenant aux sujets de fond qui ont fait couler beaucoup d'encre, en particulier les sujets relatifs à l'agriculture. Nous avons écouté les demandes du Sénat sur la réforme des chambres d'agriculture de région, qui ne pourra se faire qu'après accord de deux tiers des chambres infrarégionales. Nous avons pris en compte la demande du Sénat d'inscrire en dur les ordonnances Égalim et de faire une exception pour les produits festifs dès que le texte entrera en vigueur ; ce sera, je pense, apprécié par les professionnels alors qu'approchent

de reprendre la main sur ce texte sur la base de constats réels., c'est un texte fourni, je le reconnais volontiers, qui garde la cohérence de ses trois axes initiaux : simplification de l'administration, simplification du quotidien des Français, simplification de la vie des entreprises. Mesdames, messieurs les sénateurs, la démarche de simplification que nous prônons est concrète et doit s'inscrire dans la durée. Elle doit servir à la relance de notre pays que nous engageons en cette période de crise. Ce projet de loi, qui reflète le travail de coconstruction, contribuera à nous en donner les moyens. C'est pourquoi je vous invite à le voter. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, quoi de plus normal qu'un examen accéléré pour ce projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique ? Cela pourrait porter à plaisanterie, si ce n'était pas devenu habituel dans cet hémicycle. Hélas ! Une fois de plus, nous ne pouvons que regretter que l'exception devienne la norme. C'est d'autant plus regrettable qu'au vu du nombre d'articles ajoutés- 81 -il eût été intéressant de permettre un réexamen plus classique afin d'être pleinement au fait des dispositions que nous nous apprêtons à voter. Avoir un propos clair et synthétique sur un texte si varié n'est donc pas chose aisée. Il est difficile d'être opposé sur le principe à la simplification annoncée par ce texte. tous, dans notre quotidien, nous aspirons à cela, que ce soit dans nos relations avec l'administration, pour des travaux ou pour une simple demande de renouvellement de carte d'identité. La simplification doit être l'un des moyens permettant de redonner confiance en l'administration. Plus globalement, au regard de la période que nous traversons, je suis intimement convaincue que la relance économique, si l'on veut qu'elle soit la plus effective possible, doit être accompagnée par une simplification. Cela ne doit néanmoins pas se faire à tout prix. Si l'objectif initial de ce texte était de simplifier la vie des particuliers, la mouture finale nous donne une réalité tout autre avec une majorité de dispositions qui viennent davantage faciliter la vie des entreprises. Je pense notamment aux règles en matière de commande publique qui permettent la passation d'un marché public sans appel d'offre, quel que soit le montant, pour un motif d'intérêt général qu'il sera toujours bien difficile de qualifier. Si le relèvement des seuils de passation d'un marché public de 40 000 euros à 100 000 euros peut être bienvenu, il n'est pas une fin en soi. J'ai longtemps été maire et, chaque année, j'ai vu ce seuil être modifié pendant que nous complexifiions la commande publique en laissant les élus démunis face au contentieux que cela génère. Dans la période actuelle, notre économie aura besoin de la commande publique pour se relever et il faut noter l'intéressante disposition relative à l'accès à la commande publique pour les entreprises en redressement judiciaire introduite dans le texte. On notera aussi le passage de quinze jours à un mois du délai d'information des maires concernant les projets éoliens. C'est aussi une bonne mesure. Globalement, je suis favorable à l'ensemble des mesures venant raccourcir les délais des travaux tant que celles-ci ne viennent pas fragiliser la commande publique et sa sécurité juridique. Le constat est que, au fil du temps et de l'empilement législatif et réglementaire, le temps du papier est devenu souvent plus long que le temps du chantier. L'article 25 B ajouté par nos collègues de l'Assemblée nationale, qui supprime la soumission systématique à autorisation environnementale du plan de gestion des cours d'eau, représente en ce sens une véritable avancée en termes de gestion des milieux également d'accélérer les délais d'instruction des demandes d'autorisation environnementale pour les travaux en cas de situation d'urgence. Sur ces sujets, je regrette que nous ne soyons pas allés plus loin dans l'accélération et la simplification, mais j'espère que nous y reviendrons, notamment lors des travaux relatifs à la proposition de loi d'Henri Leroy. Au même titre, à l'article 27 , l'articulation de la procédure d'autorisation environnementale avec la procédure de dérogation concernant la directive-cadre sur l'eau nous satisfait pleinement. Néanmoins, là encore, nous faisons face à un manque de sécurité juridique concernant l'inscription de ces dérogations aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Le risque, c'est que ces nouveaux projets ne voient pas le jour faute d'inscription dans les schémas qui sont en train d'être revus et qui ne pourront être modifiés qu'à l'horizon 2027. Pour conclure, si ce texte apporte nombre de simplifications avec lesquelles nous sommes d'accord sur le fond, nous regrettons que de nombreuses dispositions n'aient pas fait l'objet d'une étude d'impact.

sur ce projet de loi dit d'accélération et de simplification de l'action publique, un projet de loi particulièrement fourre-tout, sans cohérence globale, si ce n'est la volonté de libérer l'initiative privée et de sécuriser les porteurs de projets, bref de déréguler encore et toujours au nom de l'efficacité.

L'examen en commission mixte paritaire aura d'ailleurs largement conservé le texte issu de l'Assemblée nationale : sur ces 160 articles en discussion, seulement 2 ont été retenus dans les termes proposés par le Sénat, situation que vous me permettrez de juger particulièrement déséquilibrée. Notons encore que le texte de l'Assemblée nationale s'est essentiellement étoffé à la suite de l'adoption d'amendements gouvernementaux n'ayant fait l'objet ni d'étude d'impact ni d'avis du Conseil d'État, pratique que nous jugeons particulièrement douteuse, voire inconstitutionnelle. Lors de la première lecture, nous avions voté contre ce projet de loi. Deux éléments nous paraissaient particulièrement inacceptables : la privatisation rampante de l'Office national des forêts et la régression du droit de l'environnement, notamment concernant les installations industrielles. Nous continuons de penser que, ce projet de loi ayant été déposé avant l'accident de Lubrizol, le Gouvernement aurait dû revoir sa copie, en tenant compte du résultat des enquêtes, des attentes des élus et de la population pour que plus jamais un tel accident ne puisse se reproduire. Il n'en est rien. Dans le même esprit, la seconde délibération imposée à l'Assemblée nationale à la suite de la suppression de l'article 25 portant sur les modalités de consultation du public concernant ces installations apparaît comme un véritable coup de force, pour ne pas dire un déni de démocratie. Au final, le contenu de ce projet de loi a été aggravé, notamment concernant les procédures publiques et le secret des affaires. Ce texte permet ainsi l'augmentation du nombre de marchés publics conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables, en reconnaissant une nouvelle hypothèse de dérogation lorsque « l'intérêt général » le justifie, concept bien flou à nos yeux. Nous considérons ainsi que l'intérêt général commande bien au contraire le respect des procédures afin d'éviter les conflits d'intérêts et les délits de favoritisme. Le seuil de mise en concurrence préalable et de publicité a, par ailleurs, été relevé à 100 000 euros. C'est un niveau très élevé, notamment pour les plus petites collectivités. Ces évolutions renforceront à l'évidence la défiance de nos concitoyens face aux pouvoirs publics et face aux élus. Nous estimons tout aussi inacceptable la pénalisation plus importante des squatteurs, alors qu'il y aurait tant à faire pour garantir plus efficacement le droit au logement. Comme d'habitude, vous vous attaquez aux conséquences plutôt qu'aux maux, aux faibles plutôt qu'aux puissants. L'accélération attendue par nos concitoyens n'est pas cette fuite en avant libérale, c'est celle des investissements dans les communs, alors que leur pouvoir d'achat a été grandement affecté par la crise du covid et que les bases républicaines vacillent. attendent du concret pour les mécanismes d'assurance collective, la protection de nos jeunes. Ils attendent des investissements pour l'hôpital public, pour l'école, pour la police et pour l'ensemble des services publics. Ce projet de loi, qui s'inscrit pourtant dans la démarche du grand débat ne répond à nos yeux en rien à ces urgences consacrant l'impuissance de l'État et la primauté des intérêts économiques sur les autres impératifs, qu'ils soient sociaux ou environnementaux. Pour ces raisons, nous confirmons notre vote défavorable sur ce texte.

fiction juridique a conduit le Conseil constitutionnel, dans une décision de 1999, à créer un nouvel objectif de valeur constitutionnelle : l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi.

diverses mesures du projet de loi initial n'ont qu'un lointain rapport avec la simplification de l'action publique. Ce texte constitue donc en réalité un véhicule législatif commode alors que l'agenda législatif est surchargé. Ce projet de loi, s'il ne constitue pas le grand soir annoncé lors du lancement de CAP 2022 voilà trois ans, vise néanmoins à répondre aux attentes des Français, telles qu'elles sont ressorties du grand débat national, en matière de transformation de l'action publique, publique, de simplification de leurs relations avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. La crise sanitaire et la volonté de faciliter la reprise économique rendent ces objectifs plus cruciaux encore. encore. Les travaux de notre commission spéciale ont permis d'adopter des avancées concrètes, attendues par nos concitoyens et par les entreprises, afin de simplifier nos règles, tout en préservant les équilibres de notre droit, en particulier en matière de droit de l'environnement.

en renforçant les obligations d'information des prêteurs et des assureurs. Une telle mesure concerne, mes chers collègues, près de 6 millions de particuliers, dont 80 % ignorent leur droit de changer d'assurance. Enfin, sur la thématique des squatteurs, qui a, malgré elle, donné de la visibilité à un texte qui en manquait jusqu'alors, nous avons, dans un esprit transpartisan, renforcé la procédure d'expulsion des squatteurs afin de protéger les de protéger les propriétaires et les locataires victimes de tels délits. À l'issue d'un travail parlementaire entamé en février dernier, je tiens à saluer la volonté des deux commissions spéciales, spéciales, de leurs rapporteurs et de nos deux assemblées de faire prévaloir une attitude constructive, dans le respect des apports de chacune d'elles. La convergence de vue sur la nécessité de simplifier le quotidien de nos concitoyens et de nos entreprises a permis- merci, monsieur le rapporteur -de parvenir à un bon compromis entre la Haute Assemblée et l'Assemblée Je tiens également à louer le travail considérable et remarquable des rapporteurs, ainsi que des administrateurs qui les ont assistés. Je remercie d'abord Patricia Morhet-Richaud de la qualité de son rapport, ainsi que Daniel Gremillet, qui lui a succédé,

Que serait, mes chers collègues, notre démocratie sans le bicamérisme ? », se demandait ici même, le 1 octobre dernier, le président Larcher. À cette question, je réponds que le Parlement,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, mon intervention comprendra deux points. Premier point

Positive, l'information des maires sur l'implantation d'éoliennes. Positive, la résiliation annuelle des contrats d'assurance emprunteur.

il n'en comptait que 86 au sortir du Sénat. Si je fais une soustraction, je vois, mes chers collègues, que 81 articles ont été examinés par l'Assemblée nationale et dont le Sénat n'a pas eu à connaître.

sur ce point -, nous avions adopté les nouvelles modalités du divorce au terme de la réunion d'une commission mixte paritaire, alors que le sujet avait été examiné dans une assemblée, mais pas du tout dans l'autre.

motif qu'ils n'auraient pas de rapport direct avec le texte, alors même que la Constitution prévoit que les amendements peuvent avoir avec lui un rapport indirect ? Je vous

que l'on regarde de très près en première lecture, en deuxième lecture et en nouvelle lecture, chaque mot, chaque ligne de la loi qui, souvent pendant des décennies, s'appliquera à l'ensemble du peuple français. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission spéciale, cher enfin ! -, le temps est venu d'adopter définitivement le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique, plus de six mois après que notre assemblée l'a adopté en première lecture. Du fait des circonstances que l'on connaît, son examen a été particulièrement allongé et compliqué. C'est un comble pour un texte qui vise justement à accélérer et à simplifier l'action publique ! L'essentiel est toutefois que nous puissions enfin le voter. Je me réjouis à cet égard que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord. Ce texte comporte de multiples mesures salutaires pour notre pays. pays. De nombreuses dispositions soulageront le mal français qu'est la suradministration, ce mal qui nous pousse, depuis tant d'années, tant de décennies, à soumettre tout le réel à des normes, à des réglementations, à des procédures. La suradministration étouffe tout. Elle pollue la vie de nos concitoyens, qui dépensent une énergie folle pour comprendre des règles Elle bride l'activité de nos entreprises, empêchées de produire de la valeur à cause de problèmes créés de toutes pièces par l'administration. Elle décourage aussi les élus locaux, qui craignent d'indisposer des fonctionnaires alors qu'ils devraient se consacrer tout entier à satisfaire les attentes de leurs concitoyens.

C'est l'administration qui doit servir les citoyens et les entreprises, et non l'inverse. De trop nombreuses exceptions existent aujourd'hui à ce principe, si bien qu'il n'a plus la force de la règle générale. Le pouvoir réglementaire a pris le pas sur le pouvoir législatif. Désormais, seul un tiers des procédures administratives sont effectivement soumises au principe du SVA. C'est trop peu. Il faut revenir à l'esprit de la loi et limiter le nombre d'exceptions décidées par voie réglementaire. On dit souvent que l'exception confirme la règle, mais l'excès de ces exceptions la détruit. Aussi, mes chers collègues, je vous soumettrai très prochainement une proposition de loi visant à redonner vigueur au principe du « silence gardé par l'administration vaut acceptation

voilà une bonne idée du législateur avec ce texte : nous partîmes de 50 articles, mais, par un prompt renfort, nous en vîmes 167 en arrivant au port

contribue à poursuivre le détricotage des mesures de protection de l'environnement et de la démocratie environnementale ? Des sites industriels sous-classés de manière inadaptée eu égard à leur niveau de risque échapperont au devoir de contrôle de l'État.

Des dispositions permettront de considérer les projets en cours d'instruction comme des installations existantes et d'autoriser des travaux de construction en anticipant la délivrance de l'autorisation environnementale. dispositions conduiront en fait à autoriser des installations qui pourraient se révéler non conformes dès leur premier jour de fonctionnement ou qui ne recevront pas au final toutes les autorisations

D'autres mesures visent à simplifier les démarches de fin de vie des installations industrielles soumises à déclaration. Il ne sera plus nécessaire désormais d'attester de la dépollution et de la réhabilitation de ces nouvelles friches industrielles. Quant au saucissonnage des études d'impact, il ne permettra pas de prendre en compte le cumul des différents projets et de mesurer leur impact réel sur l'environnement. prévoit de substituer une consultation électronique aux contours flous à l'enquête publique lorsque le projet soumis à autorisation ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale. Réduire ainsi le champ des enquêtes publiques constitue une régression importante en matière de démocratie environnementale. Par manque de temps, je vais moi aussi simplifier et accélérer mon intervention. Raboter les procédures environnementales et les procédures de participation du public ne permettra pas dans les faits de gagner du temps. Ce projet de loi réussit la gageure de complexifier et de déréguler en même temps. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires votera donc contre.

Le projet de loi a donc été étoffé de nombreux apports de l'Assemblée nationale comme du Sénat. Bien sûr, plusieurs concessions ont été nécessaires afin de surmonter les quelques désaccords existants entre nos deux assemblées, mais nous pouvons affirmer que le travail de concertation entre nos deux chambres a payé, et cela doit être mis en valeur. La politique, c'est aussi cela : savoir travailler en bonne intelligence avec des hommes et des femmes adversaires en politique, mais qui placent l'intérêt général avant toute chose. Très bien ! En l'occurrence, députés et sénateurs ont su s'entendre dans le but d'adopter un texte qui simplifiera la vie quotidienne de nombreux Français. Ce projet de loi, qui comprend quatre titres thématiques, contient un certain nombre de dispositifs particulièrement parlants pour nos concitoyens et pour les entreprises, parmi lesquels

plus accessible. Les personnes éligibles seront dispensées de fournir leur avis d'imposition à leur banque, laquelle s'assurera de leur éligibilité directement auprès de l'administration fiscale. Je ne reviens pas sur le droit de changer d'assurance emprunteur, nombre de mes prédécesseurs en ont parlé. Pour les entreprises, le projet de loi, dans son titre III, prévoit l'accélération des démarches afin de favoriser l'implantation d'activités dans nos territoires, sans renoncer à nos standards environnementaux. L'article 21 prévoit ainsi de renforcer la sécurisation juridique des porteurs de projets

C'est par exemple le cas du seuil de revente à perte. Sénat et Assemblée nationale sont tombés d'accord pour prolonger l'expérimentation de l'encadrement des promotions et du seuil de revente à perte jusqu'au 15 avril 2023.

administratives d'appel une compétence directe, en premier et dernier ressort, pour connaître des recours juridictionnels contre les décisions relatives aux projets d'ouvrages de prélèvement d'eau à usage d'irrigation. Cette mesure de simplification administrative,

de simplification utiles et bénéfiques pour tous. Je salue un texte qui n'a pas d'autre prétention que de rendre service aux Français et aux entreprises.

13 de ces amendements ont été retirés avant la discussion et 8 ont été déclarés irrecevables au titre de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale. Nul doute que ces dispositions nous seront ultérieurement soumises.

voter. En effet, il restait 141 articles à discuter lors de la CMP. Une centaine de ces articles ne posait pas de difficultés, le Sénat ayant même accepté de voter conforme 51 dispositions nouvelles, qui n'ont été débattues qu'à l'Assemblée nationale. très rapidement sur l'assurance emprunteur, sur laquelle Daniel Gremillet est déjà intervenu. Les dispositions qui resteront dans la loi s'inscrivent dans le droit-fil d'une proposition de loi qui avait été adoptée à l'unanimité par le Sénat en octobre 2019.

préalables à l'installation d'un parc éolien en mer introduites par l'Assemblée nationale à l'article 25 n'ont pas été remises en cause par le Sénat. Cependant, nous avons souhaité réaffirmer la prééminence des conclusions du débat public. public. Plusieurs leviers au service de la transition énergétique, en particulier s'agissant du démantèlement des installations nucléaires, du développement des installations du biogaz et de la promotion des énergies renouvelables outre-mer,

le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques

après avoir connu un long épisode économique difficile en raison de la fin des quotas et dû affronter une période de restructuration industrielle douloureuse, la filière betterave est aujourd'hui confrontée à l'une des plus grandes crises de production depuis des décennies. À la suite d'un hiver doux, une vague de pucerons a remonté la France du sud au nord, piquant les betteraves, bien avant l'arrivée des auxiliaires, notamment des coccinelles. Cela a entraîné une épidémie de jaunisse qui touche aujourd'hui près de 45 % du territoire productif français, plus particulièrement au sud et à l'est de l'Île-de-France. Les conséquences économiques pour la filière sont incontestables. Les premiers arrachages font état de baisses de rendement en moyenne en France de 15 % à 20 %- mais la moyenne n'a pas de sens en la matière -et, surtout, de baisses de rendement dans les bassins de production pouvant atteindre 50 % autour de certaines sucreries. Face au manque d'alternative efficace et au regard d'interdictions prises en 2018, la filière est aujourd'hui dans l'impasse. Les programmes de recherche ont pourtant été lancés très tôt. Ils avancent, mais n'ont pas encore abouti. Des solutions sont expérimentées, parfois depuis 2012, et sont prometteuses. Elles concernent le biocontrôle, les pratiques culturales, l'agronomie, la génétique, voire la mécanique. Aucune piste n'est écartée. L'alternative viendra vraisemblablement d'une combinaison de ces solutions. C'est ce que nous disent les experts et les scientifiques. Mais, pour la saison 2021, les producteurs sont pris de court. En attendant les alternatives,

Dans ces conditions, sans certitude que les dégâts seront maîtrisés en cas de jaunisse l'année prochaine, les planteurs réduiront légitimement leur surface betteravière. C'est le deuxième risque. Il convient de le conjurer, car cela concerne toute une filière une filière d'excellence pour la France. La betterave sucrière est une économie de proximité, en raison des difficultés de transport de la betterave. À défaut de semis et de planteurs suffisamment nombreux autour des sites d'implantation des sucreries, et faute de pouvoir faire tourner les usines plus de 100 jours, contre 50 jours attendus cette année, les risques directs de fermeture définitive sont importants. Au total, ce sont 45 000 emplois agricoles et industriels qui sont menacés. Je crois, mes chers collègues, que nous ne pouvons pas menacer de cela les Français. La fermeture de ces usines nous conduirait à terme à importer du sucre et du gel hydroalcoolique produits dans des conditions que nous refusons à nos propres producteurs au prix d'un bilan carbone nécessairement plus lourd.

qui ont investi lourdement et qui ont parié sur le gaz plutôt que sur le charbon comme les sucreries européennes concurrentes et voisines. Et le transport du champ à l'usine en France en moyenne contre 50 kilomètres en Allemagne ; cela n'est pas rien. Enfin, loin de ne servir que la filière sucrière, la pulpe de betterave représente également un apport alimentaire majeur pour nos élevages on est loin du soja OGM importé du Brésil ! C'est, par exemple, 40 % de l'alimentation du bétail dans les Hauts-de-France. Quel sens y aurait-il à sacrifier ces acquis en menaçant notre filière betteravière ? Ne manquerait-on pas de recul en sacrifiant tous ces acquis environnementaux réels, différencient, au profit d'importations accrues, y compris celles qui accentuent la déforestation au Brésil ? Analyser les risques environnementaux, et même les risques sur la santé, sur une seule des étapes de cette filière, c'est méconnaître un écosystème agricole industriel, alimentaire et non alimentaire global beaucoup plus vertueux qu'ailleurs. Il est caricatural de réduire le débat à un affrontement entre l'intérêt économique des dérogations à court terme et l'intérêt écologique de l'interdiction à long terme. Ce piège politique, très simple à caricaturer sur Twitter, nous le refusons ! Le débat oppose plutôt deux visions politiques de l'écologie. une écologie de la défiance, qui choisit d'interdire et qui conduit à une déprise de notre agriculture française, clairement observée aujourd'hui, et à une décroissance revendiquée, j'oppose ici une écologie de la confiance, parfaitement consciente de l'urgence, exigeante, mais qui s'appuie sur la réalité de nos territoires, le progrès et la recherche. Alors oui, pour toutes ces raisons, nous soutenons ce texte. Monsieur le ministre, vous avez accepté, non sans courage, de vous lancer dans ce combat. Vous aurez notre soutien, d'autant que des garanties ont été apportées par la filière et le Gouvernement. des financements supplémentaires pour la recherche sur la betterave, un plan de prévention afin de limiter l'exposition des cultures mellifères aux effets des semences utilisées à titre dérogatoire

Nous souhaiterions tous que les recherches aillent plus vite. Mais la recherche est confrontée au temps long, la recherche fondamentale comme la recherche appliquée, qui par construction est contrainte par la temporalité des saisons. Si nous sommes sûrs que les recherches avanceront d'ici à 2023, la question est de savoir si elles auront abouti

À long terme, la question de la gestion des risques sanitaires est posée. À plus court terme, c'est celle, cruciale, de l'indemnisation des planteurs et des industriels. Personne ne peut être oublié, même si cela signifie qu'il faille obtenir de l'Union européenne, à titre exceptionnel, un relèvement du plafond des aides. Il faut cependant tirer les leçons de cette crise betteravière. La première leçon est claire : il ne faut pas abandonner des filières aujourd'hui confrontées à une impasse technique. À défaut, elles disparaîtront, faute de compétitivité. Vous n'aurez pas de gains environnementaux, mais vous constaterez plus d'importations, moins d'emplois et moins de diversité agricole.

plus largement à la moutarde- notamment la moutarde de Dijon -, à l'orge ou à la carotte de Créances ... Ces produits font partie du patrimoine culinaire français, ils sont des éléments de notre flore et de nos paysages. La seule voie pour trouver des solutions

! Nous prônons l'inverse. En conclusion, mes chers collègues, la commission a voté ce texte dans un souci pragmatique d'efficacité et d'urgence. Ce projet de loi est

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a quinze ans, le Parlement réuni en Congrès votait à l'unanimité la Charte de l'environnement, un moment fort dans l'histoire politique de notre pays, qui se plaçait ainsi en précurseur pour la protection du vivant et de la biodiversité. Ce texte, comme vous le savez, a intégré le bloc de constitutionnalité à la faveur de la révision constitutionnelle du 1 mars 2005. Pourtant, le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui entre manifestement en contradiction avec la lettre et l'esprit de ce texte fondateur. Que savons-nous aujourd'hui ? Pas moins de 1 200 études démontrent que les néonicotinoïdes empoisonnent durablement les sols et tout ce qui y pousse, avec ou sans fleur, entraînant des conséquences mortifères de par leurs composés chimiques aux effets neurotoxiques graves. Ces pesticides, qui persistent pendant près de cinq ans dans les sols, peuvent contaminer les zones en bordure des champs, être transportés par ruissellement dans les cours d'eau et polluer les nappes phréatiques. Leurs effets sont tellement puissants qu'ils sont jugés 7 287 fois plus toxiques que l'ancien DDT. Depuis leur introduction dans les années 1990, la production de miel en France a été divisée par trois et la France importe plus de 70 % du miel consommé sur son sol. Cette situation est liée à la quasi-disparition des abeilles, comme en témoigne la perte de 300 000 ruches par an. Plus généralement, nous constatons aujourd'hui la disparition massive des insectes, des oiseaux, des invertébrés aquatiques et des vers de terre 80 % des insectes volants ont disparu en Europe ces trente dernières années selon une étude de 2017. Il y a même des signaux d'alarme concernant la santé humaine, selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

Au regard de ces éléments scientifiques, comment ne pas déceler la contradiction majeure entre la réintroduction de ces substances mortifères et la Charte de l'environnement ? ? Un premier considérant de la Charte affirme « que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ». Par conséquent, si rien n'est fait pour protéger la biodiversité, l'avenir de l'humanité sera en péril. Nous en avons concrètement la preuve. Si l'utilisation des pesticides, particulièrement des néonicotinoïdes, du glyphosate ou du chlordécone n'est pas totalement interdite, alors les équilibres écosystémiques seront entachés par l'empoisonnement durable du sol et du vivant. Si l'on y ajoute les dérèglements climatiques, nous sommes clairement face à un cocktail explosif pour l'avenir même du vivant. Par ailleurs, selon un deuxième considérant de la Charte, la « diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles cela signifie que mode de production et protection de l'humanité sont liés. Si le premier ne permet pas de garantir l'autre, alors les principes mêmes du développement durable ne sont pas respectés, puisque performance économique doit se conjuguer avec performance sociale et performance environnementale. Il est important de ne pas perdre de vue cette articulation. Ces considérants de la Charte de l'environnement n'instituent certes aucun droit ou liberté. Cependant, ils sont reconnus de valeur constitutionnelle par une décision de 2014 et devraient donc éclairer nos débats.

à son article 2, qui pose le principe selon lequel « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ». En réintroduisant les néonicotinoïdes, vous empêchez les agriculteurs d'exercer ce devoir, les plaçant de fait dans le rôle, non pas d'acteur de la transition écologique, mais de menace pour la biodiversité. Ainsi, vous arguez que cette exception d'interdiction est la seule voie pour permettre l'exploitation dans des conditions économiquement acceptables de la betterave à sucre. Pourtant, d'autres choix sont possibles et les alternatives n'ont été que peu étudiées. Nous noterons d'ailleurs que les cultures bio ont été moins touchées. C'est faux ! Nous considérons ainsi qu'il convient, avec le soutien des agriculteurs, d'opérer une réorientation totale de notre modèle agricole permettant de sortir du modèle des monocultures intensives. Il s'agit ainsi de promouvoir une juste rémunération, le retour des politiques du quota qui prévalaient jusqu'en 2017, la rotation des cultures et, surtout, la sortie des accords de libre-échange favorisant le moins-disant économique, social et environnemental. Je pense que vous serez d'accord Les intérêts de long terme de l'agriculture sont donc convergents avec les intérêts de préservation de l'environnement : il faut sortir du libéralisme qui exploite les hommes et gaspille les ressources pour le profit de quelques-uns. Cela n'a sous l'unique prisme de la souveraineté, comme vous le faites, monsieur le ministre, est donc en soi une méconnaissance de la Charte de l'environnement en opposant agriculture et environnement. La jurisprudence devrait, y compris sur ce terrain, vous inciter à la prudence. En effet, dans sa décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a consacré la préservation de l'environnement comme enjeu supérieur à la liberté d'entreprendre. Par ailleurs, l'article 5 de la Charte de l'environnement dispose : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. nous considérons que le principe de précaution impose de ne pas revenir sur l'interdiction générale et absolue de l'usage des néonicotinoïdes posée lors de l'examen de la loi portant reconquête de la biodiversité en 2016. de la seule et unique manière de parer à la réalisation du dommage lié à l'utilisation de ces substances incontrôlables dans l'espace et dans le temps. Ainsi, le risque grave et irréversible est largement caractérisé ; je ne reviens pas sur les études mentionnées. Par ailleurs, dans un arrêt de 2013, le Conseil d'État a jugé que l'existence d'un tel risque doit être regardée comme une « hypothèse suffisamment plausible en l'état des connaissances scientifiques pour justifier l'application du principe de précaution ». Il est clair, en l'espèce, que le risque est pour le moins « plausible » ; c'est même un euphémisme. Enfin, l'article 7 de la Charte est bafoué. Il affirme que « toute personne a le droit [ ...] d'accéder aux informations relatives à l'environnement ». Ce projet de loi, en effet, ne prévoit pas la faculté pour nos concitoyens de savoir où de telles dérogations seront accordées et quels terrains seront concernés. Enfin, et même si ce principe n'a pas à proprement parler de valeur constitutionnelle, la loi Biodiversité du 8 août 2016 a consacré le principe de non-régression du droit de l'environnement, selon lequel la protection de l'environnement ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Ce principe de non-régression est par ailleurs considéré comme un principe général du droit international de l'environnement. D'abord, au titre du principe de coopération affirmé par la déclaration de Stockholm de 1972, selon lequel les États coopèrent, non pas pour diminuer la protection de l'environnement, mais, bien au contraire, pour toujours la renforcer et « conserver, protéger et rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre Ensuite, au titre de la durabilité, qui implique un effort continuel des États pour atteindre un développement compatible avec les limites de la terre, comme cela a été réaffirmé amplement à l'occasion de la Conférence Rio+20 dans le document. Par ailleurs, le congrès le congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature a adopté, le 15 septembre 2012, une motion sur la non-régression, qui vise non seulement la nécessité de protéger les acquis de Rio, mais aussi tous les acquis des politiques et du droit de l'environnement, à l'échelle tant nationale qu'internationale. En l'espèce, permettre au pouvoir réglementaire de revenir sur une interdiction législative nous situe très clairement dans la régression environnementale. S'il est adopté, ce texte constituera un point d'appui à tous ceux qui luttent sans faille depuis 2016 pour défaire ce que le Parlement ce que le Parlement a fait. En ouvrant la brèche pour le secteur betteravier, ce projet de loi crée aussi le risque d'un contentieux sans fin pour l'ensemble des autres cultures au nom du principe d'égalité, reconnu lui aussi constitutionnellement.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, malgré ma modeste expérience sénatoriale, je dois avouer que je ne suis pas totalement surprise par le dépôt de cette motion.

et finalement assez peu de questions à trancher, hormis la date limite des dérogations, la composition du conseil de surveillance, les délais de publication des mesures réglementaires ou le spectre de ces dérogations. La volonté de nos collègues du groupe communiste républicain citoyen et écologiste d'approfondir le débat, au travers de cette motion, est donc tout à fait compréhensible. d'une part, de répondre aux interrogations liées à la constitutionnalité du texte, et, d'autre part, de prendre un peu de hauteur dans un débat sur les néonicotinoïdes où la passion prend le dessus. S'agissant de la constitutionnalité du dispositif, nos collègues estiment que ce projet de loi est « manifestement inconstitutionnel en ce qu'il méconnaît gravement plusieurs articles de la Charte de l'environnement, qui fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité depuis la révision constitutionnelle du 1 mars 2005 ». Je veux donc rappeler immédiatement l'article qui, dans la Charte de l'environnement, doit présider aux réflexions des parlementaires dans l'élaboration des politiques publiques. Il s'agit de l'article 6, Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Je ne vais l'apprendre à personne, les politiques écologiques ne se construisent pas dans un vide économique et social. Derrière chaque mesure, il y a une activité humaine, une production économique et des enjeux sociaux : c'est à l'aune de ces critères que nous devons adopter ou rejeter un texte. Chaque disposition légale et réglementaire doit être jugée à l'aune d'une analyse coût-avantage. Nous discutons ici de produits phytopharmaceutiques de la famille des néonicotinoïdes, dont il serait vain de nier l'impact sur l'environnement. Dès 2012, l'Anses a étudié le rôle des coexpositions aux pesticides et aux agents infectieux sur le phénomène de mortalité des abeilles. Petit à petit, la connaissance sur la dangerosité de ces produits a progressé et nous sommes arrivés à la situation actuelle, où seules deux substances sont autorisées au niveau européen : l'imidaclopride, uniquement pour les usages sous serre, et l'acétamipride. Concrètement, depuis 2016, 92 % des usages de néonicotinoïdes ont été éliminés. Pour certains, l'enjeu serait donc bénin, il s'agirait simplement « de finir le travail Mais c'est oublier deux éléments. D'abord, entre 2016 et 2018, l'Anses a réalisé une évaluation des alternatives chimiques et non chimiques des produits à base de néonicotinoïdes. Son expertise comporte trois volets

sait que les agriculteurs n'utilisent pas par plaisir ou par commodité des produits qui, d'une part, ont un impact sur l'environnement, et, d'autre part, représentent un coût parfois prohibitif. L'autre élément à prendre en compte pour savoir si le législateur peut venir à bout des derniers usages des néonicotinoïdes, c'est la situation actuelle de la filière betteravière. Confrontée à une recrudescence d'attaques de pucerons, celle-ci voit ses rendements diminuer de manière significative. En d'autres termes, l'absence de traitement adapté conduit à un rendement insuffisant, qui fait lui-même peser un risque sur l'emploi industriel des sucreries.

Il n'y a pas, pour la politique publique dont il est question, de solution parfaite. Soit on autorise l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique, avec les répercussions environnementales évoquées dans la littérature scientifique aujourd'hui abondante,

Surtout, cette interdiction reviendra à organiser nous-mêmes le dumping social dont nous serons victimes. Elle conduira à une perte de souveraineté, alors même que la crise du covid-19 nous a montré le caractère vital de notre autonomie alimentaire.

CO2. Pire encore, ce dumping social que nous organiserons aura une conséquence perverse directe : nous en serons réduits à importer des produits qui ne respectent pas les standards écologiques français et européens. Nous serons donc forcés de consommer des produits cultivés avec des traitements interdits en France depuis dix ans Pour toutes ces raisons, je crois que le présent projet de loi respecte l'esprit de l'article 6 de la Charte de l'environnement. Mieux encore, je pense que c'est le rejet de ce texte, et donc l'interdiction totale des produits de la famille des néonicotinoïdes, qui conduirait à méconnaître la Charte de l'environnement. C'est pourquoi le groupe Les Républicains et moi-même ne voterons pas cette motion d'exception d'irrecevabilité.

000, je le répète -, pour limiter nos importations et promouvoir un sucre produit en France dans des conditions que nous connaissons et pour sauver non seulement le sucre, mais aussi toute l'industrie agroalimentaire- le bioéthanol, la production d'alimentation pour les élevages en circuit court,

pour explication de vote. Si les arguments environnementaux font sens pour rejeter ce texte, ce dernier se heurte également à un problème juridique, qui justifie le dépôt de cette exception d'irrecevabilité par nos collègues du groupe communiste. Même notre commission des affaires économiques, majoritairement favorable à ce texte, s'est inquiétée des lacunes du dispositif, notamment d'un point de vue constitutionnel. En effet, préciser explicitement que les dérogations à l'usage des néonicotinoïdes seront réservées aux seules betteraves sucrières fait peser un risque important d'inconstitutionnalité au regard du principe d'égalité devant la loi.

Le projet de loi va également à l'encontre de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui a inscrit le principe de non-régression en tête du code de l'environnement, un principe d'ores et déjà appliqué par le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, ce qui est sidérant et surréaliste, c'est que l'on nous demande de revenir sur une disposition de cette loi qui avait par ailleurs donné une valeur législative au principe de non-régression. Je me permets de reprendre les propos de Mme la ministre de la transition écologique lors de l'examen de cette loi en 2016 : « Le texte qui vous est soumis consacre le principe de non-régression de la protection de l'environnement. Toute évolution législative future ne pourra avoir pour objectif qu'une amélioration constante de la protection de l'environnement. » Mes chers collègues, nous prenons exactement le chemin opposé ! Enfin, le projet de loi méconnaît les dispositions de la Charte de l'environnement, dont l'article 3 énonce que « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Cet article a été consacré dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel comme instituant un principe de prévention. Je rappelle- excusez du peu ! -que 1 221 études scientifiques reconnaissent la toxicité aiguë des néonicotinoïdes, ainsi que leurs modes d'action identiques sur la biodiversité- pollinisateurs, vertébrés, invertébrés. Les semences traitées avec ces substances emportent des destructions graves et irréversibles pour l'ensemble des sols et le fonctionnement des écosystèmes. Compte tenu de l'impact de ces substances sur l'environnement, permettre leur utilisation constituerait une atteinte au principe de prévention. Pour ces raisons, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires soutiendra cette motion.

monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est un sujet passionnant et passionné ! Personne ne veut des pesticides, mais vous nous proposez d'en réintroduire. Le groupe socialiste votera cette motion pour des raisons

soit il méconnaît le principe d'égalité devant la loi et emportera l'ensemble du texte dans la censure constitutionnelle ; soit il ouvre une brèche, permettant des dérogations pour toutes les cultures et remettant en cause le principe même de l'interdiction. Par ailleurs, la Commission européenne a mandaté l'Agence européenne de sécurité des aliments afin de déterminer si les autorisations d'urgence qui réintroduisent ces substances sont fondées. Sachez que, récemment, elle a rejeté les demandes de la Lituanie et de la Roumanie. Économiquement ensuite, il est tout à fait regrettable que, depuis 2016, la filière n'ait pas pu s'organiser et chercher des alternatives. Cela dit, ne la laissons pas tomber ! Monsieur le ministre, vous avez pourtant ignoré la proposition de nos collègues députés d'un plan B,

En permettant des dérogations jusqu'en 2023 et en indiquant investir seulement 7 millions d'euros dans la recherche, vous renvoyez clairement la « betterave chaude » aux calendes grecques ... Sur le plan sanitaire, comment passer sous silence les quelque 1 200 études scientifiques internationales reconnaissant la dangerosité des néonicotinoïdes. En contentant les industriels de la betterave d'un côté, vous désespérez de l'autre les apiculteurs et vous mettez en danger la biodiversité dans notre pays. Politiquement enfin, ce sujet révèle les injonctions contradictoires répétées qui règnent au sein de votre gouvernement. En 2016, Mme Pompili se réjouissait de l'interdiction des pesticides ; qu'en pense-t-elle aujourd'hui ? En 2018, le Président de la République twittait pour se féliciter de l'interdiction des pesticides tueurs d'abeilles. Monsieur le ministre, vos discours sont contradictoires : d'un côté, vous souhaitez une agriculture moins dépendante des pesticides ; de l'autre, avec ce texte, vous envoyez un signal désastreux, qui ruine la crédibilité de la parole politique en matière de changement de paradigme agricole et de lutte pour une alimentation plus saine- et c'est un agriculteur qui vous parle ! Plus globalement, ce n'est pas dans le renoncement que nous construirons un avenir alimentaire meilleur

vote. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, discuter ou ne pas discuter sur le texte qui nous est proposé au nom d'une prétendue inconstitutionnalité qui reste à démontrer est la question et indépendants, même si les avis divergent en son sein sur le fond, souhaite que nous examinions ce texte, tout ce texte, rien que ce texte. Pour cette raison, nous rejetterons cette motion.

a précisément dit : « Nous noterons d'ailleurs que les cultures bio ont été bien moins touchées ». Voilà la réalité

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, si le groupe écologiste, pourtant viscéralement attaché au débat démocratique, dépose aujourd'hui une question préalable pour rejeter unilatéralement ce texte, c'est que l'heure est grave. Depuis l'autorisation des néonicotinoïdes en France dans les années 1990 et jusqu'à leur interdiction il y a quelques années, notre pays a perdu 85 % des insectes de ses campagnes- une en moins d'un quart de siècle ! Les néonicotinoïdes ont également largement contribué à l'effondrement des populations d'invertébrés, notamment de vers de terre. Ces producteurs et ces fertilisateurs de nos sols sont aussi la ressource alimentaire de nombreux mammifères- musaraignes, hérissons, chauve-souris, etc. -et oiseaux. Imaginer leur disparition prochaine devrait toutes et tous nous plonger dans un abîme de perplexité. « La biodiversité nous concerne au premier chef, car la biodiversité c'est nous, nous et tout ce qui vit sur terre », disait Hubert Reeves. Le vivant s'effondre sous les coups de boutoir de l'activité humaine. Nous provoquons la sixième extinction de masse de l'histoire de la vie sur terre et nous continuons. Mais aujourd'hui nous n'avons plus d'excuse. Parmi les poisons que l'humanité déverse quotidiennement dans les cours d'eau, propage dans l'air ou infiltre dans les sols, les néonicotinoïdes sont l'un des plus vicieux, l'un des plus pernicieux, l'un des plus dangereux. Le plus dangereux, car il multiplie par six la mortalité des colonies d'abeilles et décime les populations de pollinisateurs.

En réalité, je ne vous apprends rien. Vous connaissez les méfaits de ces produits sur la biodiversité, vous connaissez leurs impacts sur les sols, l'eau et la vie. Vous connaissez les risques pour la santé humaine. Le débat a été tranché en 2016 et Barbara Pompili, alors secrétaire d'État chargée de la biodiversité, le disait parfaitement : « Les néonicotinoïdes sont dangereux pour notre santé, pour notre environnement, pour les cours d'eau. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas ! Imaginerait-on un gouvernement qui créerait des dérogations à l'interdiction du plomb ou de l'amiante pour les besoins de quelques industriels ? Monsieur le ministre, quelle responsabilité ! Vous savez et pourtant vous allez permettre l'utilisation d'un poison. Il a fallu vingt ans de combat acharné des apiculteurs, des écologistes, des associations, des citoyennes et des citoyens pour enfin parvenir à se débarrasser de ces pesticides. Il a fallu sept lectures parlementaires pour y parvenir, car naturellement on invoque l'urgence pour tout et n'importe quoi, mais certainement pas pour la protection de la biodiversité. Dans l'urgence la plus totale, pour faire face à une année de mauvaise récolte de betterave, pour faire face à un phénomène dont on ne sait même pas s'il se reproduira, vous voulez rouvrir la boîte de Pandore. Vous voulez introduire une dérogation scélérate dans la loi, dérogation qui ne manquera pas de faire jurisprudence et de menacer l'interdiction dans son ensemble. Car au nom du principe d'égalité devant la loi, le juge constitutionnel pourra élargir le champ des dérogations et transformer cette brèche en faille béante. Vous créez ainsi un précédent délétère que ne manquera pas d'utiliser comme exemple chaque lobby qui considérera demain que la législation écologique est un frein, ne serait-ce que léger, à ses rendements. Plus grave encore, alors que la France avait montré l'exemple en étant le premier pays à interdire les néonicotinoïdes en 2016, son renoncement annoncé est une immense victoire pour le lobby agrochimique, lui permettant de combattre l'interdiction partout dans le monde. Et le lobby écologiste ? Ce projet de loi est un cheval de Troie de Bayer-Monsanto et votre gouvernement le sait pertinemment. En baissant le pavillon, vous menacez les pollinisateurs du monde entier. Oh là là ! Pour le seul intérêt court-termiste de la filière française de sucre, vous portez un coup violent à toute la biodiversité mondiale. Quand les pesticides auront éradiqué tous les pollinisateurs et tous les vers de terre, quand nos sols seront aussi morts que les déserts de sable, quand plus rien ne poussera sans engrais chimique, alors la survie de l'humanité dépendra du pompier pyromane Bayer-Monsanto, qui aura ainsi atteint son objectif. Face à cette dystopie que l'on touche du doigt, face à cet effroyable péril, on n'attend plus ni volonté ni vision des ministres de l'agriculture du quinquennat Macron. On regrettera en revanche l'absence de la ministre de la transition écologique, dont l'action- je l'ai rappelé -avait été décisive en 2016. On la comprend : à ce niveau-là, ce n'est plus un renoncement, c'est un reniement Qu'il est loin le temps où le candidat Macron promettait l'éradication progressive des pesticides ! Trois ans après, le président Macron, incapable de tenir sa promesse sur le glyphosate portera à jamais le stigmate du retour des pesticides tueurs d'abeilles. Sacré décalage avec la réalité, avec l'attente de nos concitoyens, avec le courage de valeureux paysans comme Paul François qui, hier, gagnait définitivement son procès contre Monsanto ! Même votre majorité parlementaire assume de plus en plus mal ce décalage et plus d'un tiers des députés En Marche n'a pas voté votre Je pourrais poursuivre longtemps ce réquisitoire, mais je ne voudrais pas donner le sentiment d'égrainer les arguments d'autorité depuis un Aventin d'écologiste outragé qui mépriserait les réalités, notamment les difficultés que rencontrent les agriculteurs enfermés dans un modèle agroindustriel à l'agonie. Si nous refusons aujourd'hui ce débat, c'est que le véhicule législatif que vous nous proposez est inadapté et inepte. Nous refusons ce débat, car- nous venons d'en discuter -ce texte de loi est manifestement frappé d'inconstitutionnalité. Son étude d'impact est lacunaire, pour ne pas dire biaisée. Il est en rupture profonde avec le principe de prévention inscrit à l'article 3 de la Charte de l'environnement et avec l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de l'environnement. Nous refusons ce débat, car ce texte de loi est vraisemblablement incompatible avec le cadre européen, comme l'a souligné le 1 octobre dernier la Commission européenne, qui vérifiera la conformité de cette dérogation avec le droit communautaire. Loin de la déplorable proposition de politique agricole commune, l'Europe devrait pourtant être l'échelon adéquat pour protéger nos agriculteurs de la volatilité des cours mondiaux et engager la transition agroécologique. Au lieu de vous battre pour déroger à ses règles, vous auriez mieux fait de vous battre pour une PAC ambitieuse. Nous refusons ce débat, car nous l'avons déjà eu à de nombreuses reprises dans cet hémicycle et nous l'avons déjà tranché. La cohérence de notre Parlement est ici en jeu. Nous avons interdit les néonicotinoïdes, car c'est un poison dangereux pour la vie. Aucune étude scientifique ne vient étayer l'inverse ! Le sérieux s'impose dans cette affaire. « Il ne faut toucher à la loi que d'une main tremblante », affirmait Montesquieu, pas dans la précipitation qui guide ce débat. Nous refusons ce débat, car ce projet de loi va à l'encontre du principe de non-régression consacré par l'article L. 110-1 du code de l'environnement. La loi que nous votons n'est pas destinée à garnir les étagères poussiéreuses des bibliothèques juridiques et, là encore, nous serions avisés de respecter notre propre ouvrage. Nous refusons ce débat, car nous n'avons aucun recul sur la situation de la filière betterave à la suite de cet épisode de jaunisse. Les études de l'Anses sont en cours et la fameuse « impasse technique » n'est nullement constatée. Il conviendrait d'attendre les résultats de ces Nous refusons ce débat, car pour soutenir les agriculteurs, il aurait fallu un dispositif d'urgence pour la filière, assorti de contreparties sociales et environnementales. Avant de déroger à la loi, le cadre budgétaire aurait été un véhicule législatif nettement plus approprié, l'occasion aussi de réfléchir à un fonds important et pérenne pour les calamités agricoles. Nous refusons ce débat, car c'est une fausse réponse aux problèmes structurels de la filière betterave, qui souffre avant tout de la disparition des quotas et des pressions du libre-échange. Ainsi, malgré la jaunisse, les rendements de cette année ne seraient pas inférieurs à ce qu'ils pouvaient être au début des années 2000. Le problème, c'est qu'entre-temps la surproduction a fait s'effondrer les cours. Quand on comprendra que la surproduction agricole ne sert que la spéculation et certainement pas les agriculteurs, on pourra commencer à tenir un discours honnête et sensé. Nous refusons ce débat, car il est inepte de faire valoir les difficultés de la filière sucre, alors que l'exécutif n'a toujours pas fermé définitivement la porte au projet Sans opposition ferme et définitive de la France à ce texte, tout débat sur l'avenir de la filière est totalement vain. Nous refusons ce débat, car enfermer la filière sucre dans ce schéma délétère et à l'agonie ne rend service ni aux producteurs, ni aux industriels, ni aux ouvriers. La France est tellement en retard qu'elle est incapable de répondre à la demande nationale de sucre issue de l'agriculture biologique. Faute de pouvoir s'approvisionner en France, les détaillants bio sont obligés de se fournir au Brésil- un comble, parlait tout à l'heure de souveraineté ! Or il semblerait que la betterave cultivée en bio résisterait nettement mieux à la jaunisse. C'est faux ! Encore un bienfait de la biodiversité. Monsieur le ministre, où est le plan pour une filière française bio du sucre ? Où est votre plan pour le développement de la betterave bio ? Vous avez supprimé les aides au maintien à l'agriculture biologique, ... C'est faux ! ... cumulé les retards de paiement des aides bio et privilégié le système conventionnel. Où est votre plan pour sortir de ce modèle agricole qui détruit et asservit les femmes et les hommes ? Rien que ça ... Honteux ! N'avez-vous aucune autre perspective à offrir à nos paysans que ce piteux reniement ? Nous refusons ce débat qui méprise les apiculteurs, les arboriculteurs et tous les paysans qui dépendent de la pollinisation. Nous refusons ce débat qui ne répond qu'aux intérêts à court terme de la filière sucre au détriment de tous les autres, en particulier de ceux des paysans. Nous refusons ce débat qui est une fuite en avant criminelle. Honteux ! Nous refusons ce débat et, mes chers collègues, nous vous invitons de tout coeur à le refuser avec nous !

Mais, comme ma collègue Kristina Pluchet avant moi, je veux y voir une nouvelle possibilité de clarification. Nos collègues du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ont souhaité déposer cette motion tendant opposer la question préalable au projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières. Leur argumentaire se découpe de la manière suivante, et je ne fais ici que reprendre, scolairement, le plan de leur motion : le Parlement s'est déjà saisi de la question

S'agissant du premier élément que vous portez à notre connaissance, vous dites que « la question de l'interdiction des néonicotinoïdes a été débattue à de multiples reprises » depuis la loi d'avenir pour l'agriculture de 2014. Il y a eu, en effet, la loi biodiversité de 2016 et ses huit examens, en comptant la commission mixte paritaire, la loi Égalim ou encore la proposition de résolution relative à la préservation des insectes pollinisateurs. Selon les auteurs de la motion, une telle activité législative est en soi une raison pour ne pas légiférer davantage, surtout lorsqu'aucun élément scientifique nouveau ne vient éclairer le débat. Je vais être volontairement espiègle : si je suis votre raisonnement, une disposition légale, maintes fois modifiée pour des raisons d'agenda politique et qui se trouve matériellement inapplicable, ne pourrait pas être modifiée, au motif qu'elle l'a déjà été. Je vois dans ce raisonnement la même fragilité que celle qui a conduit à l'adoption du principe de non-régression lors de la loi Biodiversité. Je vais faire l'affront à mes collègues Philippe Bas et François-Noël Buffet de ne pas mais comment une disposition légale issue d'une loi ordinaire, et non organique, peut-elle contraindre le législateur dans l'exercice de ses prérogatives ? Il y aurait donc des lois ordinaires supérieures à d'autres ? À quoi bon, dans ce contexte, continuer d'enseigner la hiérarchie des normes à nos chers étudiants ? Pardonnez-moi cet aparté, mais c'était l'occasion de répondre au dernier grief soulevé par nos collègues du groupe écologiste sur le non-respect du principe de non-régression.

à base de néonicotinoïdes et de leurs alternatives chimiques et non chimiques, il n'y a pas eu de virage à 180 degrés dans la littérature scientifique.

Dans 39 % des cas, les alternatives chimiques reposent sur une même famille de substances actives, ou une seule substance active, voire sur un seul produit commercialisé, ce qui pose, vous l'imaginez bien, Surtout, comme l'indique le rapport, un certain nombre de méthodes potentiellement efficaces n'ont pas été retenues comme pouvant constituer une alternative pertinente aux néonicotinoïdes à l'horizon de 2020, faute d'autorisation de mise

Enfin, et c'est pour cette raison que l'interdiction avec dérogations votée en 2018 constituait une prise de risque, l'Anses évoque une difficulté à anticiper l'évolution de la pression des ravageurs en l'absence de néonicotinoïdes, quelles que soient les alternatives retenues.

Pour ces raisons, et compte tenu de la recrudescence d'attaques de pucerons, qui n'avait pas été anticipée, nous disposons d'éléments scientifiques pour étayer une telle initiative législative. S'agissant du Mercosur, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet à de nombreuses reprises. Je ne vais pas, une fois de plus, faire le procès de cet accord de libre-échange ouvrant une nouvelle voie pour le dumping environnemental, dont notre pays, nos agriculteurs et les

des collègues rappellent que la Commission européenne s'est exprimée, le 1 octobre dernier, pour préciser qu'elle entendait vérifier la conformité du présent projet de loi avec le droit communautaire, jugeant

l'argument de mes collègues ne me semble pas recevable, au motif que l'article 53 du règlement concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est sans ambiguïté : les pays membres de l'Union européenne peuvent bénéficier d'une dérogation pour ce qui concerne l'usage de ces insecticides « en raison d'un danger qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens raisonnables

Je vous invite, cher Guillaume Gontard, à vous rendre dans les champs pour observer l'infestation massive de pucerons que nous avons connue, à un stade extrêmement précoce et extrêmement inhabituel du développement de la plante, et qui a causé des ravages sans précédent.

persistant dans l'environnement. Qu'avancent les connaissances techniques du moment ? L'existence de solutions d'agroécologie, qui, visiblement, n'ont guère été sollicitées. Ce signal politique est d'autant plus désastreux que l'effondrement de la biodiversité, qui nous préoccupe tant, est aggravé par l'utilisation de ces néonicotinoïdes. Nous faisons face non seulement à un enjeu écologique, mais également à un problème de santé publique, dépassant la question de la mortalité des abeilles. À ce stade, quelques faits doivent être précisés. Les néonicotinoïdes déposés sur les semences n'y restent pas ; ils se répandent dans tout l'écosystème, et c'est là le problème ! Les études scientifiques mettent en avant les effets délétères de ces substances sur les micro-organismes, les vertébrés et les invertébrés terrestres et aquatiques. Nous savons également que les résidus obtenus après dégradation de ces insecticides peuvent être plus toxiques que les matières actives elles-mêmes. Nous observons aussi que, pour la santé humaine, il existe un lien entre une exposition répétée, même à faible dose, à ces insecticides et le développement d'anomalies cérébrales, de maladies neurologiques, voire même de cancers. C'est pour cela que ces produits ont été interdits ! Leur dangerosité a été prouvée, évaluée, mesurée, chiffrée. Regardons où nous a menés le chlordécone aux Antilles. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs

donc, à la fois, une question technique, une question économique, une question de filière. Or toutes ces questions ont été largement évacuées, par une posture idéologique qui nie complètement le débat.

ne remet en cause la toxicité des néonicotinoïdes. Mais inversement, mes chers collègues, personne ne remet en cause le fait que les pucerons ont été destructeurs cet été.

néonicotinoïdes et effondrement de la biodiversité, le lien est direct ! On nous dit d'attendre 2023, que la science va trouver des solutions. Il n'existe pas de solutions alternatives simples ! Il faut, véritablement, une évolution du modèle

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les néonicotinoïdes sont dangereux pour les humains et, en premier, pour nos agriculteurs. sont meurtriers pour les abeilles et pour l'ensemble de la biodiversité. Ils participent à la pollution et à l'appauvrissement des sols, donc à la détérioration de nos écosystèmes et du climat. C'est un fait que personne ne peut nier ! Nous avons donc fait, en 2016, un choix éclairé par la science, qui a démontré que les néonicotinoïdes sont 5 000 à 10 000 fois plus toxiques que leur ancêtre, le DDT, interdit en France depuis 1971. C'est pour cette raison que nous les avons interdits. Revenir sur cette interdiction, quatre ans plus tard, serait un échec et une régression d'un conquis environnemental. Le problème, c'est que, depuis quatre ans, aucune solution viable, respectueuse de l'environnement et de la santé publique, n'a été apportée à nos agriculteurs.

on les y a même encouragés, en leur disant que seul un modèle productiviste pourrait leur garantir un revenu décent. Cette transition écologique implique un véritable changement de paradigme, en garantissant un revenu décent et une alimentation de qualité pour toutes et tous, tout en relevant le défi

ou l'État garant de l'intérêt général, en donnant les moyens à la recherche ? Le problème réside dans le fait que les néonicotinoïdes n'ont pas été interdits dans tous les pays et, cette brèche, les industriels l'ont découverte et l'exploitent. Force est de constater, en effet, que lorsqu'il s'agit de contourner les règles environnementales, certains sont capables de développer des trésors d'ingéniosité, mais lorsqu'il faut trouver des solutions plus respectueuses de l'environnement, au vu de l'urgence climatique à laquelle nous sommes confrontés, et réfléchir à un nouveau modèle dans lequel les profits ne sont pas et ne peuvent pas être l'objectif premier, les défis leur semblent aussitôt insurmontables et les progrès sont toujours lents. Nous sommes donc face à un échec de la transition agricole et écologique depuis 2016. Mais, mes chers collègues, ne nous infligeons pas la double peine en revenant en arrière ! Que faire alors, me direz-vous ? Les pucerons existent- personne ne le nie

et, pour prévenir un autre risque, nous voulons la création d'un fonds mutuel et solidaire de gestion des risques sanitaires et climatiques, ainsi que l'introduction d'un prix plancher d'achat pour les producteurs.

Depuis 2017, la betterave a connu la fin des quotas sucriers et l'ouverture à la concurrence. Ce qui frappe le plus durement les betteraviers, ce ne sont pas les réglementations, mais bien les spéculateurs, la fin d'un marché régulé et protecteur, ainsi que le libre-échange, que vous encouragez. Exactement ! Mes

nous prenons ces décisions dans l'urgence ... Tout à fait ! ... et que, pour un certain nombre de parlementaires et de nos concitoyens, il faut se débarrasser d'une agriculture qui utilise des produits phytosanitaires comme les Français utilisent des médicaments.

gardons-nous des décisions doctrinaires et improvisées : ce gouvernement en est un peu responsable, quelquefois, mais il reconnaît ses erreurs et il sait revenir en arrière.

Je connais un certain nombre d'agriculteurs écologistes, ou qui travaillent à une agriculture plus durable, qui se retrouvent bien seuls

on ferait mieux de mobiliser davantage d'énergie pour trouver des produits de substitution et de nouvelles méthodes productives.

De ce que le Parlement décidera au sujet de ce texte dépendront en effet les prochaines réponses du Gouvernement aux filières en difficulté. C'est sûr ! C'est une solution sans coût budgétaire que nous propose en l'espèce le Gouvernement. d'une réponse bien tentante, à l'heure où l'État doit soutenir de nombreux secteurs face aux conséquences économiques de la covid-19. En outre, cette réponse évite au Gouvernement d'avoir à se pencher sur les causes profondes de la crise que traverse la filière betteravière française. La détresse de cette dernière doit être entendue. Mais avant de prendre une telle décision, lourde de conséquences- nous le savons tous -, nous devons nous poser les bonnes questions. Premièrement, une dérogation à l'interdiction de l'usage des néonicotinoïdes résoudra-t-elle durablement les difficultés de la filière ? Non, puisque les causes profondes sont d'ordre systémique. Certes, la jaunisse de la betterave exacerbe les difficultés des producteurs dans certains territoires, mais elle est loin d'expliquer à elle seule la fragilité de la filière sucrière. En 2019 déjà, les principaux sucriers fermaient des usines et supprimaient des emplois ; c'était non pas le contrecoup d'un déficit de production de betteraves, mais la conséquence directe de la suppression, en 2017, des quotas sucriers et du prix minimal garanti, qui a entraîné un effondrement des prix. En 2016, les acteurs de la filière betterave espéraient que la libéralisation du marché du sucre leur permettrait d'augmenter leurs rendements et leurs marges : tel n'a pas été le résultat, bien au contraire. Aujourd'hui, ils pensent que la réintroduction des néonicotinoïdes permettra de sortir leur filière de l'ornière. Pourtant, la filière a surtout besoin que le législateur soit à ses côtés pour l'accompagner vers une plus grande résilience. Deuxièmement, l'autorisation d'utiliser ces substances dangereuses résoudra-t-elle le problème de la campagne de 2020 ? Évidemment non,

usages autorisés des néonicotinoïdes étudiés n'ont pas permis de trouver de solution de substitution, et les betteraves n'en faisaient pas partie. La filière betterave-sucre elle-même voit désormais une issue à cette impasse. Ainsi, le 2 octobre dernier, elle a remis au ministre de l'agriculture

Non, mille fois non : nous avons déjà pris trop de retard face à l'urgence environnementale, au-delà de la seule question climatique. La biodiversité est tout aussi menacée par les activités humaines : un million d'espèces animales ou végétales sont menacées d'extinction, soit une espèce sur huit Plus personne n'ignore le rôle joué par les insectes pollinisateurs dans la préservation de cette biodiversité. Plus personne n'ignore non plus le rôle des néonicotinoïdes dans la disparition des abeilles. L'Union nationale de l'apiculture française, l'UNAF, estime ainsi que 300 000 ruches sont anéanties chaque année à cause des néonicotinoïdes- d'où leur surnom « tueurs d'abeilles ». Pour nous rassurer, le Gouvernement avance que les plants de betteraves ne produisent pas de fleurs mellifères. Mais les fleurs ne sont pas la seule source de mellification, sinon il n'y aurait pas de miel de sapin

Si le Gouvernement veut vraiment aider cette filière, il ne doit faire l'économie ni d'un soutien financier de court terme ni d'une réflexion de fond sur sa structuration. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain fera, dès l'examen du projet de loi de finances, des propositions pour la création d'un fonds d'urgence permettant à la filière de passer le cap de la campagne de 2020.

ce projet de loi est une réponse d'urgence pour sauver notre filière betteravière, qui est aujourd'hui en grande difficulté. Il autorise l'utilisation des néonicotinoïdes par enrobage de semences

La France est le premier producteur européen de sucre. Cette filière compte 46 000 emplois et 21 sucreries. Elle est aujourd'hui durement frappée par la jaunisse, qui touche tous les modes de production et tous les territoires.

Mes chers collègues, l'enjeu est essentiel : il y va de notre souveraineté alimentaire et de notre autonomie de production. La dérogation que nous examinons aujourd'hui est prévue par le droit européen.

tel choix nous contraindrait inévitablement à importer des produits dont les normes environnementales et sanitaires sont souvent moins strictes que les nôtres. Par ailleurs, il est important de rappeler que, pour 2020, notre excédent d'échanges agroalimentaires continue de reculer de plus d'une centaine de millions d'euros. Gardons à l'esprit que la filière betterave représente plus de 1 milliard d'euros d'excédent commercial. L'utilisation des néonicotinoïdes en enrobage sur la betterave, plante non mellifère, est à ce jour la seule solution efficace à court terme. Permettez-moi de revenir quelques instants sur l'historique de cette interdiction d'utilisation. Elle a été adoptée en 2016. Force est de constater qu'elle est entrée en vigueur en 2018 sans qu'aucune solution de substitution ait été prévue ou même étudiée. Comme disait Talleyrand : « Quand il est urgent, c'est déjà trop tard. Une étude d'impact aurait permis de constater que cette interdiction n'était pas réalisable dans un tel laps de temps. Je souhaite vivement qu'à l'avenir l'on rende les études d'impact systématiques,

La dérogation proposée est strictement encadrée dans le temps, jusqu'en 2023. D'ici là, nos meilleurs alliés seront la recherche et l'innovation, lesquelles sont indispensables pour promouvoir le plus grand nombre Les réponses devront être multiples ; la recherche génétique semble la plus prometteuse, et elle devra être combinée à d'autres solutions. Par ailleurs, je souligne le travail accompli par la filière sucrière, afin de rechercher des solutions pour les pollinisateurs, particulièrement avec les producteurs de luzerne. Les pollinisateurs sont les meilleurs alliés des agriculteurs : il faut que nous fassions la promotion de solutions adaptées à leur protection. Précisément, le dispositif est strictement encadré pour protéger la biodiversité parmi les seule l'utilisation l'enrobage des semences sera autorisée. Je salue la limitation à 2023 de cette dérogation et l'interdiction temporaire de plantation et de replantation de végétaux mellifères. Je considère qu'un minimum de deux années s'impose pour une rémanence maîtrisée.

que nos deux assemblées s'accordent rapidement, afin que ces dispositions entrent au plus vite en vigueur. Ce projet de loi est encadré et proportionné. Il est absolument nécessaire. C'est pourquoi les élus du groupe Les Indépendants voteront majoritairement pour, en appelant toutefois

Ce qui ne nous convient pas, c'est un modèle qui broie un certain nombre de paysans depuis trop longtemps. L'interdiction des néonicotinoïdes, obtenue après vingt ans d'une lutte lancée par les apiculteurs, était l'une des trop rares avancées des dernières années dans le combat contre les pesticides. Elle est aujourd'hui mise à mal par un texte qui non seulement permet de répandre de nouveau des poisons dans l'environnement, mais envoie un signal désastreux quant à la volonté des pouvoirs publics d'amorcer réellement la transition agroécologique de l'agriculture. Pourtant, d'autres solutions existent, et elles sont nombreuses : réduction de la taille des parcelles ; semis plus tardifs ; jachères favorisant la présence d'auxiliaires des cultures ; rotations longues

Les témoignages d'agriculteurs engagés dans des systèmes alternatifs le montrent : il est possible de mettre en oeuvre des solutions agronomiques pour se passer de ces molécules. Des scientifiques l'affirment également.

de faire face à l'urgence des pertes économiques de la filière. Pour cela, nous proposons la mise en place de mécanismes écoconditionnés, qui pourraient coupler aides publiques et fonds de mutualisation- nous y reviendrons lors de l'examen

C'est la fuite en avant d'un modèle industriel à bout de souffle qui provoque ces difficultés techniques. Des sols presque morts, des cultures sous perfusion d'intrants, un environnement appauvri au point que les ravageurs n'ont plus aucun prédateur de nouveau les néonicotinoïdes, c'est alimenter ce cercle vicieux. On le sait, la crise de la betterave est avant tout liée à la dérégulation des marchés, depuis la fin des quotas en 2016. Nous devons, au contraire, travailler à un commerce international équitable et permettre une véritable relocalisation de l'alimentation. Ce serait aussi l'occasion de favoriser l'émergence d'une filière de production de sucre bio, dont la France s'honorerait d'être le leader.

Alors que nous sommes dans une situation d'urgence, la décision que nous prenons aujourd'hui est perçue comme un souffle pour raviver le feu. Allons-nous continuer ainsi jusqu'au dernier souffle ?

Ces agriculteurs sont en première ligne depuis le début de la crise sanitaire pour nous permettre de manger, tout simplement. Avant tout, je tiens donc à leur rendre un vibrant hommage. J'étais vendredi à Haussy, petite commune de l'arrondissement de Cambrai, avec Hélène Levrez et son mari, agriculteurs betteraviers. Ils me disaient : « L'agriculture, c'est un métier de passionné.

J'ai pu le vérifier en parcourant, ces dernières semaines, les routes de mon département et en échangeant avec celles et ceux qui font notre alimentation. Dans le Cambraisis, le Solesmois, le Dunkerquois ou la Pévèle Carembault, j'ai rencontré des agriculteurs betteraviers confrontés à une situation tout à fait exceptionnelle, même si je sais que le département du Nord n'est pas celui qui paye le plus lourd tribut au virus de la jaunisse. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Nous parlons d'un texte qui n'a d'autre ambition- mais n'est-ce pas là la plus belle d'entre toutes, celle qui doit animer nos actes ? -que d'aller vers l'idéal et de comprendre le réel.

Une seule solution s'offre à nous, au-delà des anathèmes de toute nature qui inondent nos boîtes aux lettres électroniques et qui n'ont d'autre objet que de stigmatiser celles et ceux qui voteraient pour ce texte, au nom de la préservation de la biodiversité.

Pour moi, pour beaucoup d'entre nous, la transition écologique consiste à mettre en cohérence les temps de la politique, de la science et de l'agriculture avec la loi de la nature ; mais l'analyse du passé ne résoudra pas, à elle seule, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Oui, ce projet de loi vise à mettre rapidement un terme à l'usage des néonicotinoïdes sans pour autant sacrifier les filières et la protection de l'environnement. Je rappellerai donc ce qu'il est et, surtout, ce qu'il n'est pas. Ce projet de loi n'est pas une autorisation de mise sur le marché. Il n'introduit pas davantage l'utilisation d'un nouveau pesticide : il met un terme à l'usage des néonicotinoïdes. Je le dis fermement, car il faut que les choses soient claires pour tout le monde : ce texte n'encourage pas l'agriculture française à revenir aux pesticides, bien au contraire.

Ce projet de loi permettra donc d'en finir avec les derniers 8 % qui embarrassent la filière de la betterave. Cet effort mérite toute notre attention : mobilisons les moyens d'accompagnement nécessaires au lieu de laisser cette culture souveraine sur le bas-côté, comme le souhaitent nombre de détracteurs politiques. Nous nous devons de relever le défi du virage écologique et d'une agriculture durable et pérenne. C'est ce virage que nous prenons et que nous encourageons à suivre. Ce texte ne s'oppose en rien à une telle vision de la société et les adaptations qui lui ont été apportées ne le réduiront pas à un chèque en blanc. Il garantit que, pendant trois ans, notre agriculture se focalisera sur la fin des néonicotinoïdes. Il garantit que, dans nos territoires, nous aurons toujours des champs de betteraves pour alimenter des sucreries. M. le ministre l'a rappelé : il y va de notre souveraineté économique et alimentaire, et, me semble-t-il, de notre capacité à accélérer la transition agroécologique. Ce projet de loi ne constitue pas non plus une régression pour le droit de l'environnement, ce qui serait, bien entendu, inconstitutionnel. Il s'inscrit dans le droit européen en vigueur et prolonge le régime d'interdiction qui était le nôtre depuis 2018, avec des possibilités de déroger strictement encadrées. D'un point de vue social, il s'agit surtout de ne pas tuer des exploitations betteravières et de ne pas jeter au chômage des femmes et des hommes qui travaillent dur, depuis des années, dans l'espoir, souvent, de transmettre leur exploitation aux générations futures. Ce texte ne vient pas d'en haut : il émane de nos territoires ruraux. Enfin, ce débat n'oppose aucunement les « pro » et « anti » néonicotinoïdes, pour la bonne et simple raison que nous tous, ici, faisons partie de la seconde catégorie. Oh ! Personne ne nie les dangers de cette substance, ni le Gouvernement ni moi-même. Les acteurs de la filière ne considèrent pas davantage les néonicotinoïdes comme une solution durable : tous souhaitent en sortir. Le recours aux néonicotinoïdes est, en l'occurrence, une solution d'urgence. C'est le seul moyen de faire face à une situation intenable pour la filière betteravière et sucrière. Souhaitons-nous conserver notre place de leader européen ou la laisser à d'autres par dogmatisme, pour ensuite compenser cette perte de leadership par l'importation de sucres étrangers dont la production ne respecte pas nos critères environnementaux ? L'égoïsme écologique du « plus vert que vert chez moi et tant pis pour les autres » ne résoudra pas les problèmes. Les auditions menées par nos deux rapporteurs l'ont clairement montré : la sortie des néonicotinoïdes passera non pas par une solution unique, mais par la combinaison de plusieurs évolutions. d'entre elles relèvent d'un changement de pratiques culturales, et de culture au sens large, qui doit conduire à repenser la question des équilibres au sein des parcelles en favorisant l'installation d'auxiliaires naturels prédateurs des pucerons, ainsi que de bandes enherbées et de haies. Nous sommes toutes et tous bien persuadés de la nécessité de « remettre de la complexité » dans les parcelles. C'est cette complexité que je vous invite à assumer aujourd'hui : je suis convaincu que la situation à laquelle nous faisons face ne trouvera de solution apaisée que par le dialogue, le respect mutuel et le refus des positions dogmatiques.

Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire », a dit un jour Georges Clemenceau. Nous voulons tous ici faire de l'agroécologie une réalité, mais nous sommes confrontés à une crise sans précédent ... Il faut vraiment conclure, cher collègue ! Nous le disons et, en votant ce texte, nous le faisons, avec courage et détermination

un métier qui recouvre tous les enjeux actuels de notre planète : l'indépendance alimentaire, le maintien de la biodiversité, la santé publique, les emplois non délocalisables, l'aménagement du territoire.

Nous reconnaissons tous la nocivité de ces produits. Je l'ai dit plusieurs fois dans cette enceinte, nos votes doivent tenir compte d'un équilibre fondamental entre les trois axes qui découlent de l'agriculture : l'économie, l'environnement et la santé. Bien souvent, nous privilégions un axe par rapport à un autre. Là est notre erreur, car tout est question d'équilibre, tout est question de raison. S'agissant de la méthode, revenir sur une loi est une faute, car cela entraîne, une fois de plus, un déficit de crédibilité : les citoyens ne veulent plus de ces tergiversations.

conjoncturelle- une attaque exceptionnelle de pucerons sur les betteraves -et une situation structurelle- la crise de la filière sucrière depuis plusieurs années. Quel est le contexte ? La production du sucre dans le monde se partage essentiellement entre le sucre de canne, pour 79 %, et le sucre de betterave.

les restructurations en bio restent faibles par rapport aux autres filières. Parmi les dérogations, l'Allemagne, partenaire essentiel européen, a choisi les néonicotinoïdes par pulvérisation plutôt que par enrobage,

il faut que votre gouvernement soutienne cette filière par des aides conditionnées à la pratique d'une agriculture durable ; il faut enfin profiter du plan de relance pour aider la transition économique de la filière et ainsi l'inscrire dans la pérennité.

chers collègues, nous devons soutenir cette filière, mais pas en prenant des décisions qui n'auront aucun effet sur la pérennité de ses entreprises. Nous devons prendre des décisions en conscience et en responsabilité, avec les professionnels qui nous permettent de rester leader en Europe et toujours placés au niveau mondial.

Madame la présidente,

J'ai eu trop souvent à dénoncer leur incompréhension du monde agricole, ainsi qu'un manque de clairvoyance et de réalisme. Aujourd'hui, je dois reconnaître, monsieur le ministre, que ce sentiment change à votre égard. Je veux même Je veux même vous remercier d'avoir eu le courage de reconnaître et de corriger une erreur collective sur les néonicotinoïdes. les néonicotinoïdes. Cette erreur a bien été collective- oui, collective -, car d'un côté, on trouvait tous ceux qui, par des incantations, ont voulu faire un exemple de leur détermination à supprimer toute molécule chimique de l'agriculture, sans se poser aucune question-

l'autre côté, se tenaient tous ceux qui voulaient y croire et jouer le jeu, avec l'envie de faire toujours mieux en pensant que le progrès allait à lui seul apporter la solution.

à ce moment-là, certains tiraient déjà la sonnette d'alarme en prédisant ce qui allait se passer et ce que nous avons vécu, sans jamais avoir été entendus. Vous avez eu le courage, monsieur le ministre, de reconnaître reconnaître l'étendue des dégâts sur la culture de la betterave sucrière, qui avoisinent parfois 70 % dans certaines zones ; le courage de reconnaître que le remède est pire que le mal, quand on fait jusqu'à huit traitements curatifs,

sachant que cette disparition sera amplifiée par le manque de compétitivité française face à nos concurrents allemands ou brésiliens. Ne l'oublions pas, en effet, notre économie est concurrentielle et mondialisée.

même si l'on sait que, dans ce domaine, le temps est souvent très long. Il ne faudrait pas que le délai de trois ans que vous avez proposé soit insuffisant ; attention à ne pas reproduire la même erreur qu'en 2016. Corriger avec bon sens, c'est aussi corriger rapidement, comme vous le faites. Le temps presse : les semis de betterave de 2021 se décident maintenant. Sans cette évolution, le choix des agriculteurs se limiterait à semer pour ne rien récolter ou, carrément, à laisser tomber cette culture pour assurer la pérennité de leur exploitation. Tout cela devrait nous servir de leçon pour l'avenir. Nous ne devrions plus prendre une décision d'interdiction en nous laissant seulement guider par le dogmatisme, sans avoir auparavant constaté et assuré la crédibilité des alternatives techniques. Je ne comprends pas que les adeptes de la formule « il est interdit d'interdire », tous ces bien-pensants, qui sont d'ailleurs souvent ceux-là mêmes qui nous demandent de nombreuses expertises, des démonstrations, qui nous imposent une multitude d'exigences, de rapports en tout genre, n'appliquent pas la même formule pour ces sujets.

Dans ce cas précis, le produit concerné permet tout d'abord le maintien de la santé économique de la filière sucrière française, qui contribue chaque année à plus de 1 milliard d'euros d'excédents dans la balance commerciale.

devra tout faire pour favoriser la croissance. La betterave sucrière pourra continuer à y contribuer pleinement. Ce ratio permet aussi le maintien de notre autonomie alimentaire.

Je vous rappelle le rapport que j'ai réalisé en 2019, lequel met en évidence que plus d'un jour et demi par semaine

La leçon, c'est aussi de savoir retrouver de l'objectivité, de la raison et de la modération. Notre agriculture n'a pas à être clouée au pilori ; elle a su, pendant des décennies, se servir de l'innovation, de la recherche, du progrès technique pour évoluer, pour s'améliorer, pour se perfectionner. Monsieur le ministre, je proposerai, lors de l'examen du projet de loi de finances, une évolution importante du budget de la recherche, ne soyons plus contraints de revenir sur des décisions prises à l'emporte-pièce, en mettant en oeuvre, avant la prise de décision, des méthodes intelligentes qui nous permettraient de sortir de l'écologie punitive et d'entrer dans l'ère de l'écologie constructive, en adéquation avec le bien-être de nos agriculteurs, la réalité du monde économique et de l'évolution de notre planète. À ce sujet, il est essentiel de garder à l'esprit que le nombre d'habitants sur Terre est passé de 2,5 milliards

Si nous ne prenons pas suffisamment en compte cette évolution de la population et les risques de migration qu'elle pourrait imposer, le résultat de tous les efforts que nous aurons faits pendant des années pourrait s'écrouler du jour au lendemain, alors que l'agriculture et la production de denrées alimentaires seront cruciales pour l'équilibre du monde et pour le maintien d'une France forte, capable de nourrir son peuple. Au-delà de la réintroduction des néonicotinoïdes, monsieur le ministre, nous devons nous poser les bonnes questions

Républicains vous soutiendra dans cette démarche, comme il le fera aujourd'hui sur ce projet de loi. La

L'expansion de la maladie de la jaunisse risque de tuer ce fleuron de notre agriculture : il faut réagir ! C'est l'objet de ce projet de loi, qui permet de déroger jusqu'en 2023 à l'interdiction de l'utilisation de produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes.

la maladie de la jaunisse altère la physiologie des plantes en entraînant une réduction quantitative des récoltes et qualitative du taux de sucre de la betterave. Depuis le 1 septembre 2018, date d'interdiction des néonicotinoïdes, il a fallu recourir à des méthodes alternatives, mais celles-ci ne sont pas du tout à la hauteur du problème et parfois même, leurs conséquences sur l'environnement sont encore plus significatives. L'Anses, elle-même, reconnaît que les indicateurs de risque alimentaire des néonicotinoïdes sont inférieurs à ceux des solutions alternatives. Il faut donc continuer à chercher le bon substitut, mais nous sommes dans l'urgence, dans le présent, et nos territoires ruraux déjà fortement affectés par la crise économique appellent à l'aide, car cette filière se trouve clairement dans une situation d'impasse technique. Le ministère de l'agriculture annonce que la perte de rendement s'élève en moyenne à 13 %. Dans certains départements, les pertes se situent entre 40 % et 50 %, ce qui se traduit économiquement par une perte supérieure à 1 000 euros par hectare.

Que vont faire les planteurs des zones les plus touchées ? C'est simple, ils renonceront demain à semer de nouveau ce type de produits, sauf s'ils obtiennent la garantie de ne plus supporter les mêmes difficultés. Au-delà des fermetures de sites de production que nous avons déjà eu à subir, notamment dans mon département, la Somme, en raison de l'arrêt des quotas, c'est la fin d'une souveraineté économique nationale, déjà bien altérée, qui est délibérément programmée si nous ne réagissons pas. Un plan social massif devra alors être élaboré pour accompagner les 46 000 emplois directs et indirects de cette filière, car les incidences du recul de la production du sucre affecteront, vous le savez, nos industries agroalimentaires, chimiques, pharmaceutiques et, naturellement, les industries liées à la production du carburant alternatif éthanol, pour lequel je me suis tant battu dans une autre chambre parlementaire. Je rappelle, alors que l'on parle de relocaliser les productions de souveraineté sanitaire, que c'est cette filière qui produit également le gel hydroalcoolique, si essentiel pour lutter contre l'épidémie du moment. Bref, ce n'est pas un combat contre l'indispensable évolution des pratiques agricoles, c'est un appel à la raison et un cri du coeur pour sauver un pan entier de notre économie nationale, déjà si malmenée. Avec 445 000 hectares plantés et 38 millions de tonnes produites, la France est le premier producteur de sucre de betterave européen et le deuxième mondial. Nous en sommes fiers. Il est crucial pour cette filière, qui regroupe 25 000 agriculteurs et vingt et une sucreries, qu'elle obtienne la même dérogation que celle dont bénéficient déjà douze États membres de l'Union européenne, comme l'Allemagne, la Belgique, ou encore la Pologne. est l'objet de ce projet de loi, lequel, en s'appuyant sur l'article 53 de la réglementation européenne, autorise l'usage de ces produits l'enrobage des semences, à l'exclusion, bien sûr, de toute pulvérisation. le groupe Union Centriste vous invite à soutenir ce texte, qui répond à trois urgences : ne pas laisser l'industrie entière s'effondrer, soutenir intelligemment dans le temps une transition agroécologique prometteuse et, enfin, préserver notre agriculture et notre souveraineté économique nationale.

Quatre années se sont écoulées sans que la filière de la betterave sucrière ait mis en place de solutions alternatives durables d'agroécologie. Quatre ans après le vote de 2016, rien n'a été fait pour assurer le succès des décisions politiques volontaristes et courageuses prises pour le bénéfice de tous, la France était précurseur, qu'elle avait entraîné l'Union européenne dans son sillage vertueux. Ainsi, vous vous dérobez à la première difficulté d'une filière, comme s'il n'y avait rien d'autre à faire que de renoncer. En réponse à cette crise, vous faites le choix d'une certaine facilité. Nous ne partageons pas les solutions économiquement court-termistes et écologiquement désastreuses que vous proposez. Celles-ci nous opposent dans notre rapport à l'environnement, à la biodiversité, à l'économie et à la santé elles marquent aussi une véritable fracture politique entre des choix soumis à la pression des lobbies, dévastateurs d'un point de vue écologique, et notre ferme volonté de poursuivre les engagements que nous avons pris en 2016 pour l'environnement. Une nouvelle fois, vous privilégiez l'économie au préjudice de l'écologie. Les effets délétères des néonicotinoïdes n'échappent pourtant à personne dans cet hémicycle ; nous connaissons la neurotoxicité de ces molécules et leurs conséquences sur les écosystèmes et le vivant ; nous savons que ces insecticides prennent une large part dans la chute inexorable de la biodiversité. Oui, les espèces sont menacées. D'ailleurs, la Cour des comptes européenne relève les échecs des actions menées et les fortes sommes engagées pour enrayer le déclin de la biodiversité, sans effet. C'est grave : nous n'arrivons pas à arrêter ce terrible déclin, c'est un fait, et c'est là le véritable problème

Dans ce contexte, ce projet de loi fait fi de la science, va à contre-courant de l'évolution de la société. C'est un échec écologique fracassant, un non-sens environnemental qui va à l'encontre du droit de l'environnement et menace directement notre santé. Un intérêt général d'ordre supérieur devrait pourtant s'imposer à nous, celui des biens communs l'eau, l'air, la terre, la nature en somme qui, dans son ensemble, nous offre et nous rend tellement de services, gracieusement. En retour, vous lui offrez la réintroduction d'une substance 7 000 fois plus toxique que le DDT les colonies d'abeilles sont décimées- 37 % au sein de l'Union européenne, tout de même. Or les abeilles sont des lanceuses d'alerte, leur santé est un véritable indicateur de l'ensemble de la chaîne des pollinisateurs sauvages et, plus largement, des insectes. Sans leur présence, la pollinisation, pourtant indispensable à la production agricole, serait compromise.

pour atteindre les lacs et les rivières. Le néonicotinoïde y persistera des années durant, constituant une pollution de l'eau que nous consommons. La plante, quant à elle, sera entièrement irriguée d'une sève toxique et deviendra un végétal pesticide. Ainsi, c'est l'ensemble de la chaîne du vivant qui est menacée. Le monde bruissant, chatoyant et foisonnant de la nature est d'une magnifique complexité ; les interactions y sont variées et complexes, elles forment des écosystèmes à l'équilibre insoupçonné, que l'on découvre parfois alors qu'il est déjà trop tard. Ce texte offre, enfin, le spectacle d'un revirement politique : vous mettez fin non seulement aux mesures adoptées en 2016, mais aussi à celles de 2018, prises dans le cadre de la loi Égalim, qui élargissait l'interdiction des néonicotinoïdes. Drôle de temporalité, alors que la France s'apprête- ou

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à saluer tout d'abord l'excellente et pertinente analyse de notre collègue Sophie Primas, rapporteur de ce projet de loi.

Le comble est que cela est dû à un refus de la part de l'État français de prendre ses armes ! Nous vous remercions, monsieur le ministre, de votre lucidité conduit à accepter cette réadaptation de nos pratiques agricoles jusqu'en 2023, le temps que des solutions de substitution, de traitement compatible avec la protection de l'environnement, soient trouvées. Faisons confiance à la recherche Nos agriculteurs n'attendent que cela, car ils sont aujourd'hui stigmatisés, ils sont traités de criminels de la nature, de tueurs d'abeilles,

Ce dogme est terrible, car il stigmatise, il donne des leçons, il mène des procès d'intention : d'un côté, il y aurait les vertueux, les protecteurs, les bien-pensants, les partisans d'une agriculture saine, bio, écolo de l'autre, les irresponsables, les destructeurs, les mauvais esprits, partisans de la malbouffe chargée de polluants, de conservateurs et de colorants. Non, le modèle agricole que nous souhaitons tous est plus complexe, plus difficile à cerner il consiste à concilier l'activité économique, la survie d'une filière avec les impératifs de développement durable, l'économie et l'écologie. Je rappelle que, dans mon département, la fermeture de la sucrerie de Bourdon a entraîné la suppression de près de cinquante emplois. Ce projet de loi tend à répondre à cette conciliation, je dirais même qu'il permet une réconciliation de la réalité et de l'idéal, car il n'y a pas d'idéal sans réalisme. l'idéal n'est pas l'idéologie, laquelle stigmatise, attaque, réduit le champ des possibles et, surtout, ignore la réalité et la rend dangereuse pour le quotidien de nos citoyens. Aussi, il faut faire confiance à l'esprit de responsabilité de nos agriculteurs et à l'intelligence et au bon sens de nos paysans. Très bien ! Ceux-ci souhaitent faire confiance à l'écologie positive et non punitive : depuis les premiers rapports de l'Anses, les produits phytopharmaceutiques ne sont pas considérés comme des tueurs d'abeilles à eux seuls. On ne peut, certes, ignorer leur part de responsabilité, mais ils n'expliquent pas à eux seuls la mise en danger des pollinisateurs ; plusieurs facteurs concomitants doivent être pris en considération si l'on veut apporter des solutions efficientes. Par ailleurs, nos idéologues anti-agriculteurs conventionnels affirment haut et fort que des solutions de substitution existent déjà.

Je me demande, mes chers collègues, ce que cherchent les « ultraverts » qui nous harcèlent, voire nous menacent, sur les réseaux sociaux, nous donnent des leçons de morale, nous accusent de ne pas penser à l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants ; je leur réponds que je n'ai pas de leçon de morale à recevoir et que je n'accepte pas les procès d'intention ! Bravo ! Je leur réponds que, pour mes enfants et mes petits-enfants, je suis fier de défendre l'emploi de la filière agricole je suis fier de défendre une agriculture nourricière, surtout en ces temps de pandémie ; je suis fier de faire confiance à la recherche de mon pays pour une économie de croissance, et non de décroissance je suis fier de préserver les intérêts de nos paysans français face à la concurrence déloyale ; enfin, je suis fier de défendre nos paysans vertueux, premiers aménageurs de nos territoires et premiers écologistes de France. Excellent

le Conseil constitutionnel, « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ». Dans ce cadre, le Conseil constitutionnel a déjà jugé qu'il y avait un intérêt général à soutenir une activité économique déterminée et identifiée comme stratégique ou en difficulté, et que cela

mais la réussir avec la filière française ! La discussion générale est close. Mes chers collègues par courrier en date de ce jour, M. le Premier ministre a informé M. le président du Sénat que le Gouvernement ferait, jeudi 29 octobre 2020 après-midi, une déclaration suivie d'un débat et d'un vote, en application de l'article 50-1 de la Constitution, relative à l'évolution de la situation sanitaire et aux mesures nécessaires pour y répondre. Les modalités d'organisation du débat à la suite de la déclaration du Gouvernement seront définies par la conférence des présidents qui se réunira demain, à En conséquence, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande que l'examen du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur

heures trente : déclaration du Gouvernement, en application de l'article 50-1 de la Constitution, suivi d'un débat et d'un vote puis, l'après-midi et le soir : projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses dispositions de gestion de la crise sanitaire Vendredi 30 octobre 2020 au matin : suite du projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, puis suite du projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche pour les années 2021 à 2030

où les hautes cheminées de briques des sucreries dominent les plaines du Noyonnais, du Compiégnois, du Beauvaisis, du plateau picard et d'Estrées-Saint-Denis. Devenue terroir sucrier, notamment après que Napoléon eut imposé le boycott de l'importation du sucre de canne, qui enrichissait la perfide Albion, l'Oise, à l'instar de nombreux départements français, a vu son activité agricole faire une large place à la culture betteravière. Certes, la modernisation et la concentration ont entraîné la fermeture de bien des sucreries ; mais l'activité reste importante et fait vivre de nombreuses familles- il suffit de circuler dans nos campagnes en ce moment pour voir les norias de poids lourds et autres engins en action. Mais jusqu'à quand ? Si nous n'instaurons pas cette dérogation, strictement encadrée et temporaire, non seulement nous condamnons nos betteraviers, mais nous ne sauvons pas pour autant la planète et les générations futures. En effet, nous continuerons à consommer du sucre « néonicotinoïdé », produit par nos voisins belges ou allemands ou même bien plus loin, au Brésil, avec une traçabilité et une pureté bien aléatoires ... Étrange vertu écologique schizophrène, qui nous verrait sacrifier sciemment nos planteurs au bénéfice de leurs concurrents, défendus, eux,

ailleurs, des effets économiques à long terme de la chute des populations de pollinisateurs sur les productions agricoles qui en ont besoin pour assurer leur rendement ? met en garde contre de futures famines, faudra-t-il, comme en Chine, polliniser à la main les cerisiers ? Pourquoi céder à la facilité et aux pressions de différents groupes, au lieu de proposer des alternatives d'ordre économique, agronomique et technique pour aider les acteurs à supporter le risque sur leur parcelle et à faire évoluer leurs pratiques agricoles pour lutter contre le virus de la jaunisse ? Il y a des solutions ! Nous avons rencontré de nombreux agriculteurs biologiques qui cultivent de la betterave

Pour tous ceux qui sont aujourd'hui malades d'un cancer, pour tous ceux qui souffrent parce qu'ils ont perdu l'un des leurs, pour toutes les associations qui ont déposé de multiples

de Victoire Jasmin, je veux réagir à la communication du Gouvernement sur ce projet de loi, qui nous paraît problématique. Ces dérogations nous sont présentées comme une fatalité, une solution proposée à contrecoeur, mais nécessaire pour la souveraineté alimentaire.

Or, ce qui nous est proposé, c'est une dérogation sur l'enrobage des semences. En d'autres termes, avant même de connaître la situation sanitaire des plantations de betteraves, le Gouvernement autorise ces produits en préventif sur plus de 400 000 hectares En effet, au moment de la mise en production des semences et de leur plantation, il sera encore trop tôt pour estimer correctement le risque de jaunisse. Cette utilisation des néonicotinoïdes est donc tout sauf ciblée et limitée

Le modèle choisi par notre voisin repose donc sur le refus de tout traitement préventif de l'ensemble des surfaces de betteraves et sur l'autorisation- uniquement si les conditions de l'émergence de pucerons sont réunies -de l'acétamipride. Les quantités de néonicotinoïdes répandues dans l'environnement sont alors bien moindres. Je n'entends pas faire l'apologie de la pulvérisation, dont les inconvénients sont majeurs. Je tiens à souligner que l'enrobage des semences n'est en rien plus écologique

Je vous trouve le ministre d'un gouvernement attentiste et pas du tout prospectif. Il y a eu une véritable paresse dans ce domaine. Où est le courage, monsieur le ministre ? On vous dit courageux ; je suis plus qu'interrogatif. Le courage et l'audace, c'est d'accompagner l'agriculture vers des filières de qualité, respectueuses de l'environnement et rémunératrices. Le courage et l'audace, c'est de protéger notre agriculture des insupportables distorsions de concurrence devant nos avancées

monsieur le ministre, je ne le trouve pas. Cette loi est véritablement régressive ; elle ne fera que creuser le fossé entre l'agriculture et nos concitoyens. La parole est à M. Fabien Gay,

la production de betteraves est consacrée aux biocarburants. On pourrait faire évoluer ce taux. Vous parlez de souveraineté alimentaire : interrogeons-nous sur la souveraineté alimentaire de l'Europe en matière de sucre bio.

Pendant six années, je n'ai eu de cesse de plaider pour le renforcement de la recherche et de l'innovation. Ce projet de loi revient sur une loi qui a interdit il y a quelque temps l'usage de molécules qui ont un nom imprononçable. Ce projet de loi est un retour en arrière. Ce projet de loi est un pas de clerc. Ce projet de loi est la consécration d'un échec. Ce projet de loi préfigure le scénario qui se produira pour le glyphosate. Ce projet de loi préfigure que les objectifs et les ambitions des rois de la transition écologique sont accompagnés de moyens de mendiants. Je ne voterai pas pour un échec. Je ne voterai pas pour donner de faux espoirs. Je m'abstiendrai, car je ne veux pas entrer dans un débat qui n'est qu'un sparadrap.

Je suis convaincue que l'activité betteravière de notre pays souffre davantage aujourd'hui du capitalisme que des parasites et des pucerons dont nous parlons depuis tout à l'heure. Comme l'a rappelé mon collègue du Puy-de-Dôme, Jean-Marc Boyer, le groupe sucrier Cristal Union a fermé plusieurs sucreries en France, dont celle de Bourdon à Aulnat. Résultat : 350 emplois directs et indirects ont été supprimés, 300 planteurs ont vu leur activité betteravière affaiblie et, pour certains, totalement arrêtée. Cela prouve une fois encore que seuls les grands groupes industriels tirent les ficelles en vue de la rentabilité sans se soucier des femmes et des hommes qui composent ce corps de métier et des conséquences sur leur vie.

porté ces messages et que vous n'avez pas financé suffisamment les alternatives que nous sommes aujourd'hui dans cette situation. On aurait pu collectivement accepter une tuile- la jaunisse du puceron -, mettre sur la table les indemnisations pour passer ce mauvais moment et sauver la filière. C'est tout à fait possible : l'État l'a souvent fait face à des calamités agricoles. Au lieu de ça, nous revenons en arrière,

Ne dites pas qu'il y aurait ceux qui connaissent l'agriculture et qui défendent les agriculteurs et ceux qui ne le feraient pas. Ce n'est pas digne de ce débat.

des avancées importantes pour mieux protéger la biodiversité et pour lutter contre la disparition des insectes pollinisateurs, notamment les abeilles, qui sont indispensables aux plantes, aux cultures et à la vie et qui permettent une meilleure préservation de notre environnement.

Comment pourrait-on aujourd'hui régresser sur ces enjeux majeurs, alors même que tout le monde s'inquiète de l'avenir de la planète ? C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, je voterai contre la réintroduction des néonicotinoïdes. La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn,

question très difficile, car si nous sommes tous concernés par l'environnement, par les générations futures et par la protection de notre santé, nous sommes aussi tous concernés par les agriculteurs, qui sont des aménageurs et d'ailleurs

générale, qu'on fait un amalgame entre la crise structurelle de la filière et la crise conjoncturelle causée par cette maladie provoquée par les pucerons.

Mais si ! Nous avons aujourd'hui une culture qui pourrait bénéficier d'un traitement pour subsister. Nous avons tous été choqués

Lors de leur audition, les agriculteurs nous ont assuré que derrière des cultures de betteraves il n'y avait jamais de cultures de plantes mellifères, mais des cultures de céréales, de blé et d'escourgeon pendant un, voire deux

Si vous acceptez cette dérogation pour les betteraviers, monsieur le ministre, que répondrez-vous à la filière noisette, à la filière maïs et à d'autres encore ? Vous nous engagez dans une voie de renégociation permanente avec toutes les filières agricoles concernées par les semences enrobées. Vous défendez, ici même, au Sénat, les arguments des agrolobbies, qui pourront à leur tour se prévaloir d'un discours gouvernemental assumé devant la représentation nationale.

prévoyait l'interdiction des néonicotinoïdes en 2020. Je n'épiloguerai pas : l'agenda gouvernemental est tel qu'il lui était sans doute impossible de venir que la politique environnementale s'en trouve sérieusement altérée, tout au moins dans ses symboles et dans sa réalité. En avez-vous bien évalué l'impact environnemental ? N'y avait-il pas d'autre solution que cet aménagement législatif privilégié par le Gouvernement dans une attitude que je qualifierai de court-termiste ? On aurait pu soutenir financièrement la filière de la betterave grâce au plan de relance et l'accompagner dans la transition qu'elle n'a pas faite d'elle-même. Au lieu de ça, vous nous proposez, par ce texte,

En 2016, comme simple citoyen, j'ai suivi les débats parlementaires qui ont abouti à l'interdiction des néonicotinoïdes. Aujourd'hui, nouveau sénateur, il me semble entendre les mêmes objections, les mêmes arguments, les mêmes protestations sur les désastres économiques et sociaux, les mêmes demandes de dérogation très dérogatoires et les mêmes incantations à l'égard de la recherche de nouveaux produits chimiques Tout cela a déjà été entendu et surmonté par la loi de 2016. Alors, ne régressons pas ! Les néonicotinoïdes sont indiscutablement des poisons redoutables pour la faune et la flore.

en aurait aussi sur d'autres filières agricoles et sur d'autres réalités économiques comme les apiculteurs et les producteurs de colza ou de tournesol, dont les rendements baissent quand les pollinisateurs disparaissent. Face aux mêmes enjeux,

une dérogation de même nature. Elle opte plutôt- cela a été rappelé -pour du curatif ciblé sur les seules superficies touchées. C'est un moindre mal marqué du sens de la mesure auquel appelait

de néonicotinoïdes pour les betteraves sucrières. Je regrette que les abeilles et les pollinisateurs ne soient pas au centre des débats. Je regrette le peu d'intérêt pour d'autres productions en souffrance

Les lobbies sont effectivement moins puissants pour la production fruitière. Je regrette- cela a été rappelé par un collègue sénateur LR -le manque de moyens de l'Inrae afin d'avoir enfin, pour des productions comme les betteraves et certains fruits, une recherche qui trouve. Je voterai donc contre cette loi de dérogation, qui vise à prolonger l'utilisation des néonicotinoïdes enrobés et à rester dans l'impasse. Je protège aussi l'égalité entre agriculteurs, qui ne sont pas traités de la même manière selon leur production et leur région. C'est une rupture d'égalité. Je regrette enfin que certains collègues s'appuient sur les exemples allemand et belge pour dire que nous devons faire pareil et déroger. C'est une façon singulière de considérer l'Europe. En liberté, en conscience, je voterai contre ce texte, car rien n'a avancé depuis 2016, et je crains que, si nous ne mettons pas chacun au pied du mur et devant ses responsabilités, rien ne bouge. Dans trois ans, nous aurons, hélas, les mêmes débats et les mêmes résultats. La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte,

Bonhomme, sur l'article. Certains ont regretté le débat excessivement simplifié qui prenait un tour un peu caricatural. Peut-être faut-il partir de la réalité qui s'obstine et qui contrevient parfois aux lectures dogmatiques.

Arrêtons de croire possible une alternative issue de la substitution d'un produit chimique par un autre produit chimique. La recherche ne va pas aussi vite que la destruction du vivant ; elle n'apportera pas de solution miracle si le perdure. La conjoncture n'est pas exceptionnelle ; elle se reproduira et se reproduit déjà. La monoculture, soutenue par les néonicotinoïdes, appartient au passé. Elle a tout gâché : les insectes, les sols, les cours d'eau, la vie des travailleurs de la terre. Ce sont ces pratiques que nous devons reconstruire au lieu de nous arc-bouter sur un modèle agricole dépassé. Il est clair que toutes les avancées en matière de biodiversité ou de stratégie bas-carbone entraîneront des difficultés réelles et transitoires. Prévoir ces difficultés en accompagnant ces secteurs dans leur conversion plutôt que de déroger à ces engagements au moindre coup de vent défavorable est ce que nous attendons d'un gouvernement qui nous paraît plus adepte d'une écologie du dire que d'une écologie du faire.

Soyons sérieux ! Nous en sommes, aujourd'hui, à prendre une décision qui engage notre pays, et nous n'avons pas le droit de nous tromper. Je vous remercie de bien vouloir le comprendre

n'avons pas attendu qu'il y ait un problème pour nous pencher sur l'évolution de nos méthodes agriculturales

Ne cassons pas aujourd'hui une transition qui ne peut pas se faire du jour au lendemain, au risque de faire sauter toute une agriculture et toute une économie. Il faut un peu de temps pour n'avons pas attendu qu'il y ait le premier débat au Parlement pour y travailler. Nous y travaillons, ne nous laissez pas au milieu du champ.

Malheureusement, ce n'est pas en disant que nous comprenons le problème et que nous appelons à une alternative que nous sortirons cette filière de l'ornière, précisément parce que l'alternative n'existe pas.

Toutefois, tous ceux qui ont pratiqué des dispositifs de biosécurité savent à quel point c'est compliqué, puisqu'il faut que la vitesse de propagation de la coccinelle dépasse celle de propagation

pas que je suis le ministre de l'agrochimie ou, madame Rossignol, n'en appelez pas aux générations futures. Je prends cette décision en tant que ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en tant qu'ingénieur agronome et en tant que père de quatre enfants. Monsieur